J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur le projet de loi de finances rectificative pour 2019 est parvenue à l'adoption d'un texte commun. Monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, l'ordre du jour appelle les réponses à des questions d'actualité au Gouvernement.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, un pont s'est effondré lundi à Mirepoix-sur-Tarn, dans mon département. Mes premières pensées, auxquelles j'associe mes collègues de Haute-Garonne, vont, bien évidemment, aux familles des deux victimes de ce drame. L'heure n'est pas aux polémiques. Il est trop tôt pour incriminer qui que ce soit, même si les circonstances de cet accident semblent maintenant connues. Triste coïncidence, ce drame intervient six mois après la publication du rapport de la mission d'information sur la sécurité des ponts, présidée par Hervé Maurey. Notre pays compte plus de 200 000 ponts ; 90 % d'entre eux sont gérés par les collectivités locales. Parmi eux, 25 000 sont d'ores et déjà répertoriés comme étant en mauvais état structurel. La situation est particulièrement inquiétante pour les 100 000 ponts qui relèvent des communes ou des intercommunalités.

Ce rapport très pertinent préconise de mettre en oeuvre un véritable plan Marshall pour les ponts, en créant un fonds d'aide aux collectivités. Comme on l'a fait pour les tunnels après la catastrophe du Mont-Blanc, avec la mise en place de moyens importants pour les sécuriser, il faut aujourd'hui débloquer des crédits

À quand un accompagnement adapté, urgent et nécessaire, pour les communes et les intercommunalités qui n'ont pas les moyens financiers, techniques et humains requis pour assurer, seules, la sécurité de ces ouvrages ?

vous avez rappelé le drame survenu avant-hier matin à Mirepoix-sur-Tarn ; je veux à mon tour avoir une pensée pour les victimes et leurs familles, pour les services de secours, qui se sont mobilisés très tôt, et pour certains des témoins du drame, qui ont eu le courage de porter assistance aux personnes alors en péril.

très rapidement d'un carnet de santé de l'ensemble des ponts et les doter de capteurs permettant de surveiller leur état en temps réel. Sur ce sujet, monsieur le sénateur, soyez assuré de la mobilisation de l'État, qui partage votre ambition en la

La parole est à M. Bernard Cazeau, pour le groupe La République En Marche. Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Mme la ministre des solidarités et de la santé. Aujourd'hui, l'hôpital est malade, mais il est vrai que cela vient de loin. L'hôpital n'a pas supporté les évolutions successives qui lui ont été infligées depuis plusieurs années, tant en matière financière que pour son sans parler de l'exercice médical de ville, qui a beaucoup évolué depuis vingt ans et dont la pratique est, à mon avis, en partie responsable de l'engorgement des urgences.

madame la ministre, en conférence de presse, ce matin, M. le Premier ministre et vous-même avez apporté une réponse forte, concrète et rapidement applicable, qui permet de faire face à l'urgence. Elle s'articule autour d'une accélération de la stratégie « Ma santé 2022 » et donne suite aux demandes des professionnels de santé à travers trois mesures phares.

une valorisation financière des équipes engagées, à hauteur d'environ 300 euros, ou encore une revalorisation des métiers d'aide-soignant.

En quoi les décisions prises par le Gouvernement nous permettent-elles d'espérer que, demain, l'hôpital va jouer le rôle fondamental qu'attendent les Français ?

il nous a fallu prendre la mesure de cette crise légitime et, surtout, proposer des solutions nouvelles qui répondent aux attentes. Transformer le système de soins, tel était l'objectif de la stratégie « Ma santé 2022 ». Nous avons engagé cette réforme afin de replacer le patient au coeur du système de privilégier la qualité des soins, plutôt que des logiques comptables. Ce plan visait à réorganiser la médecine de ville et à réarmer les hôpitaux de proximité, afin d'assurer la continuité des soins pour nos concitoyens. C'est également le sens du pacte de refondation des urgences, qui vise à éviter des passages inutiles dans les services d'urgences en réorientant les patients qui peuvent être pris en charge ailleurs. Enfin,

Cette réforme vise aussi à assouplir le fonctionnement des hôpitaux : nous faisons confiance aux responsables de terrain et nous voulons faciliter les prises de décisions. Enfin, la réforme présentée par M. le Premier ministre vise à redonner des moyens

dans la vie locale et à la proximité de l'action publique. Ce texte, que le Sénat a adopté à l'unanimité moins deux voix, vise à remettre la maire au centre de la gouvernance locale, alors que de nombreux élus font part de leur désarroi. Certains sondages indiquent même que seul un maire sur deux envisagerait de se représenter. Nous ne dirons jamais assez combien le mandat de maire constitue la quintessence de la vie démocratique, le coeur battant de notre République. Le Président de la République l'a d'ailleurs rappelé hier dans son hommage aux maires de France. Vous le savez bien, madame la ministre, le Sénat a beaucoup travaillé pour aboutir à un texte d'équilibre, ce dont votre collègue Sébastien Lecornu, qui était chargé de représenter le

», l'assouplissement de l'intercommunalité, les indemnités des élus ou encore la territorialisation des compétences intercommunales facultatives. M. Lecornu l'a dit lui-même : l'une des ambitions de ce texte, que vous avez voulu coproduire avec le Sénat, est de répondre au sentiment de dépossession des élus, en particulier face à la complexité normative. C'est ce que notre Assemblée a souhaité faire en introduisant davantage de proximité et de souplesse dans la gouvernance des collectivités, et en remettant la commune au coeur du pacte républicain pour redonner du sens, du contenu, de l'attrait et des moyens au mandat de maire.

On aurait pu aussi imaginer une concertation des partenaires sociaux, voire un Grenelle de l'hôpital ! Rien de tout cela : votre mépris du Parlement et des corps intermédiaires n'est pas nouveau, mais sa violence continue de nous heurter. Il y a un an, votre méthode a été exactement la même pour répondre aux « gilets jaunes Vous ne réagissez que quand la colère sociale vient enrayer la mécanique de votre machine néolibérale qui broie, jour après jour, le service public. Après avoir minimisé les problèmes, après avoir louvoyé, il vous aura fallu plus de huit mois de mouvement social pour commencer à mesurer la gravité de la situation, mais comme d'habitude, vous faites le service minimum ! Vous reprenez une partie de la dette ; c'était indispensable. On rappellera que ce sont les règles européennes qui obligent les hôpitaux à se financer auprès des banques privées : une aberration Pour revaloriser les salaires, pour embaucher, pour soulager les personnels et éviter les fermetures de lits, le monde hospitalier vous demande de doubler l'objectif national de dépenses de l'assurance maladie, soit une augmentation de 4 à 5 milliards d'euros par an. Vous proposez dix fois moins ! Sur les augmentations de salaire, rien Sur l'ouverture de lits, rien ! Sur les embauches, rien ! Sur les internes, rien non plus ! Ce que vous concédez d'une main avec des primes insuffisantes, pour certaines catégories de personnel seulement, vous le reprendrez demain avec la réforme des retraites. Nous ne pouvons donc pas imaginer que votre réponse soit exhaustive. Monsieur le Premier ministre, merci de nous préciser les autres mesures que vous envisagez pour répondre à la crise hospitalière !

Des agents mieux traités et des conditions de travail améliorées, ce sont des patients mieux accueillis et mieux soignés dans des lieux plus adaptés. Nous donnons également à chaque hôpital une plus grande marge de manoeuvre financière, comme ils le demandaient. Nous dégageons 1,5 milliard d'euros sur trois ans : c'est autant d'argent supplémentaire pour recruter, pour moderniser, pour ouvrir des lits là où il en faut. Les établissements auront l'autonomie nécessaire pour investir, parce que nous la leur donnons, mais aussi parce que nous allons les soulager financièrement du poids de leur dette, à hauteur d'un tiers de la dette des hôpitaux, soit 10 milliards d'euros sur trois ans. Enfin, nous nous sommes engagés à ce que les tarifs des hôpitaux, c'est-à-dire les prix qu'ils facturent à l'assurance maladie, et qui représentent une grande partie de leur budget, non seulement ne baissent plus, contrairement à ce qui s'est passé jusqu'en 2018, mais augmentent

tout cela sera rendu aux établissements de santé. Je l'ai dit et je le répète : je veux que les hôpitaux bénéficient directement de toutes les économies réalisées par une meilleure programmation et une meilleure pertinence des soins. Nous devons tout cela aux agents hospitaliers : ils attendaient ces annonces, qui sont à la hauteur de leurs espérances ! La parole

alors les retraités, les chômeurs, les précaires, les étudiants, les pompiers, les personnels de santé, les cheminots, les « gilets jaunes » et tout le peuple que vous mettez à l'agonie finiront par vous les ouvrir ! L'hiver social arrive et il sera rude

Mme la secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie évoquait, le 5 novembre dernier, la volonté du Gouvernement d'engager une réforme des impôts de production, accusés de « grever les finances des entreprises ». Cette idée, probablement soufflée par le Medef, résonne de plus en plus au sein de votre ministère,

Après la suppression de la taxe professionnelle et, plus près de nous, le tour de passe-passe de la taxe d'habitation, c'est tout simplement la décentralisation que vous continuez de détricoter. Ce coup de canif fiscal « économique » ne ferait en effet que dégrader l'autonomie fiscale de nos collectivités ; par voie de conséquence, il affaiblirait les services rendus aux usagers. En effet, ce sont les élus locaux qui, jour après jour, doivent répondre aux attentes légitimes de leurs administrés ; ce sont ces élus locaux qui oeuvrent, jour après jour, pour garantir le développement harmonieux et solidaire d'un village, d'une ville, d'un département, ou d'une région, tout simplement pour construire une République des territoires qui soit plus juste ! À l'heure des mouvements sociaux- « gilets jaunes », étudiants, blouses blanches, policiers, agriculteurs, enseignants -, au moment où la République aurait plutôt besoin de se rassembler, vous ne trouvez rien de mieux à faire que de poursuivre cette entreprise de démolition de la fiscalité locale, en mettant cette fois-ci la CFE et la CVAE dans votre viseur. Très bien ! Nous savons tous que, dans une démocratie, l'impôt est un lien de citoyenneté. Il est donc de notre responsabilité de lui redonner toute sa légitimité, en veillant à ce qu'il soit réparti équitablement, dans le respect de la justice sociale. Et ce n'est pas en le supprimant, monsieur le ministre, que vous apporterez plus d'équité. Ma question est simple. Les maires sont réunis en ce moment en congrès, à la porte de Versailles. Pouvez-vous leur affirmer que cette petite musique qui consisterait à inscrire dans une trajectoire de baisse la CFE et la CVAE va enfin s'arrêter de jouer ?

garantir, comme j'ai déjà eu l'occasion de le faire, de même que M. le Premier ministre à plusieurs reprises, à l'ensemble des élus de France que la suppression de la taxe d'habitation, qui est avant tout une mesure de justice fiscale et de pouvoir d'achat pour nos compatriotes, sera intégralement compensée aux collectivités, non par des dotations, comme cela a toujours été le cas, mais, à l'euro près, par des recettes fiscales dynamiques et pérennes, pérennes, de manière à ce que l'autonomie financière des collectivités soit assurée et à ce qu'on ne reproduise pas les travers du Fonds national de garantie individuelle des ressources, qui avait été mis en place à l'occasion de la suppression de la taxe professionnelle, de manière aussi à ce que les collectivités ne connaissent pas à nouveau, comme cela a toujours été le cas, un amoindrissement des allocations de compensation, que l'État cesse toujours de verser à un moment ou à un autre. Nous changeons de modèle, nous faisons en sorte que la compensation soit intégrale, durable et, surtout, dynamique. Je pense que nous pourrons, les uns et les autres, nous accorder sur ce sujet.

Nous pouvons aussi ouvrir un certain nombre de chantiers sans nécessairement poser la question du niveau des ressources. Les barèmes de la CFE sont-ils toujours satisfaisants pour les élus ? Je ne le crois pas. Les recettes de la CVAE sont-elles toujours prévisibles pour les collectivités ? Ce n'est pas le cas non plus ; toutes celles et tous ceux qui ont une expérience intercommunale ont pu le mesurer. Peut-on progresser, comme cela a été le cas de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels ? Oui, et il faut continuer ce travail de « sincérisation ». Nous avons un objectif : faire en sorte que le panier fiscal sur lequel s'appuient les collectivités soit stable, qu'il soit juste et qu'il soit durable ! La parole est à Mme Colette Mélot, pour le groupe Les Indépendants

des accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH). La loi pour une école de la confiance a favorisé la valorisation de leur statut, en transformant les contrats aidés en CDD de trois ans. En outre, 4 500 postes supplémentaires ont été déployés, portant le nombre d'accompagnants à 90 000. Nous savons que le taux de scolarisation de ces enfants s'est considérablement amélioré. En deux ans, 40 000 enfants supplémentaires ont été accueillis en milieu scolaire ordinaire, portant ces effectifs à 361 500. En dépit de ces avancées, que nous saluons, la scolarisation des enfants handicapés reste un défi pour le Gouvernement et un problème quotidien pour les familles qui n'ont pas encore de solution. Les associations témoignent du fossé entre les annonces et la réalité. Ils seraient 11 000 enfants à ne pouvoir bénéficier de l'accompagnement nécessaire, faute de moyens déployés et faute d'attractivité du métier d'accompagnant. Le Président de la République a fait de la scolarisation des élèves en situation de handicap une priorité du quinquennat. Le Gouvernement se donne trois ans pour bâtir le socle de l'école inclusive et assurer à chaque élève un égal accès à l'éducation, selon ses besoins particuliers. Monsieur le ministre, à l'heure de la mobilisation nationale des accompagnants d'élèves en situation de handicap, quelle réponse d'urgence proposez-vous aux 11 000 élèves sans solution ? Quelles actions pour améliorer concrètement les conditions de travail des AESH, qui n'ont pas tous bénéficié des mesures annoncées ?

Il leur a rendu hommage- le contraire aurait surpris -, mais il a laissé le chantier de l'acte III de la décentralisation en jachère, sans rien annoncer de neuf. Or les nuages s'accumulent sur les libertés locales. La recentralisation est en marche, qui place les communes sous la dépendance de l'État et déresponsabilise les élus. L'autonomie financière recule avec l'usine à gaz de la compensation de la taxe d'habitation. Les dotations s'érodent, car elles ne sont pas indexées sur l'inflation. Les subventions discrétionnaires des préfets sont préférées à la dotation d'investissement, qui seule est libre d'emploi. À travers les « contrats de Cahors », l'État s'immisce dans la libre administration des collectivités. Il oppose aussi une fin de non-recevoir au rééquilibrage des relations entre communes et intercommunalités. Rien n'est fait pour faire obstacle au communautarisme. Sur ce point, on sait maintenant ce que le Président de la République ne veut pas, même si on ne sait toujours pas ce qu'il veut. Monsieur le Premier ministre, allez-vous prendre la pleine mesure de ces réalités et des menaces d'asphyxie qui pèsent sur la démocratie locale ?

vous avez brossé un tableau bien noir de la réalité vécue par les maires. Après tout, pour reprendre votre formule, il aurait été surprenant qu'il en soit autrement !

tout cas comme cela que, pour ma part, je le regarderais -, on voit très clairement une période où, pendant trois ans, les dotations ont baissé,

C'est parfaitement documenté. Vous savez très bien que nous avons décidé de ne pas nous engager dans un big-bang périmétrique pour remodifier les répartitions de compétences, lesquelles avaient

nous allons finir de remplacer la taxe d'habitation par une recette fiscale dynamique, dans le cadre d'un dispositif, qui, comme l'a remarquablement expliqué M. le secrétaire d'État voilà quelques minutes, garantit aux communes des ressources pérennes.

de l'Association des maires de France lui-même qui nous a fortement invités à ce que, sur les projets relatifs à la décentralisation, sans mettre la question à l'écart,

ira bien plus loin que tout ce qui a été fait jusqu'à présent en matière de différenciation. Comme vous êtes un homme qui croit à la réalité des faits plutôt qu'aux promesses, monsieur le président Bas, je vous renvoie à ce que nous avons fait pour l'Alsace

pour la réplique. Monsieur le Premier ministre Philippe, je vous l'accorde : il y a eu pire que votre gouvernement. Voyez-vous, la commune n'est pas une nostalgie. Les maires ne sont pas des faire-valoir. Ils n'ont que faire des flatteries. Ils appartiennent à la démocratie du concret. Ce ne sont pas des marchands de bonheur.

En effet, la semaine dernière, pendant l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, en présence de Mme Buzyn, le Président de la République a annoncé que des réformes de l'hôpital seraient annoncées par M. le Premier ministre lui-même.

convaincant. Les professionnels de santé attendaient un plan de sauvetage, ils n'ont eu que du rafistolage. Les revalorisations se sont transformées en primes ponctuelles, soumises à conditions. Les 300 millions d'euros de plus pour 2020 sont à mettre en perspective avec les 800 millions d'euros de déficit annuel des hôpitaux. Après avoir contribué à endetter les hôpitaux, faute de leur donner les moyens de fonctionner, vous vous contentez d'alléger leur dette d'un tiers. Monsieur le Premier ministre, vous nous avez présenté le plan « Ma santé 2022 » il y a quatorze le plan pour les urgences il y a six mois. Manifestement, ils n'ont pas atteint leur objectif. On peut malheureusement d'ores et déjà parier qu'il en sera de même pour vos dernières annonces. Monsieur le Premier ministre, pourquoi n'avez-vous pas fait le choix d'une réforme en profondeur de l'hôpital ?

vous m'interrogez sur le plan que, ce matin, Mme la ministre des solidarités et de la santé et moi-même avons présenté. Un mot d'abord pour dire ce qui motive ce plan au-delà de ce décrochage et de ce sentiment d'abandon parfois exprimé par toute une série de professionnels qui font vivre l'hôpital public : une régulation budgétaire terrible dans les dix dernières années, une transformation de la gouvernance à l'intérieur de l'hôpital qui a éloigné les médecins des lieux de décisions, une réforme profonde de l'organisation territoriale qui a donné le tournis à l'hôpital public. Ajoutez à cela les 35 heures

de discours ! Ces décisions ont conduit l'hôpital public à une situation dont on pourrait dire, si on était dans l'aéronautique, qu'elle relève presque du décrochage.

pour qu'il puisse passer cette phase de transformations indispensables, qui a été décrite par Mme la ministre dans le cadre du plan « Ma santé 2022 ». J'observe- et je suis certain que vous l'observez également, -que, dans les manifestations et remarques exprimées par les corps intermédiaires auxquels vous comme moi sommes attachés, on n'entend pas la contestation des orientations qui ont été fixées par Mme la ministre dans le cadre du plan « Ma santé 2022 ». Vous le savez parfaitement. Il y a, au contraire, une forme d'adhésion, mais

parce qu'il y a urgence. Tel est le sens du plan d'action que nous avons présenté ce matin, qui n'est pas un petit plan d'action, puisqu'il s'agit de mettre sur la table, pour les trois ans qui viennent, 1,5 milliard d'euros

a été divisé par deux et, dans la même période, l'endettement de l'hôpital public a crû de 40 %. Ce phénomène rend les hôpitaux publics insusceptibles de dégager les marges de manoeuvre qui leur permettent d'envisager leur avenir. C'est précisément la raison pour laquelle, à côté de ces 1,5 milliard d'euros, plus les 450 millions d'euros, nous avons décidé d'opérer une reprise de dette. Je n'ai pas le souvenir, mais je parle sous votre contrôle, monsieur le président Milon, qu'une telle reprise de dette ait été couramment réalisée dans le cadre de l'hôpital public : 10 milliards d'euros de dettes en trois ans, c'est massif. 10 milliards d'euros de dettes en trois ans, c'est massif. Cela permet, compte tenu des taux d'intérêt, de dégager à terme, c'est-à-dire au bout des trois ans et de la reprise, environ 800 millions d'euros de marge de manoeuvre pour les hôpitaux. C'est considérable. C'est considérable. Il ne s'agit pas simplement de moyens, il s'agit de remettre en avant l'attractivité de l'hôpital public par des primes- c'est vrai -, par la mise

Ce plan d'action renforcé, ce plan d'urgence, a vocation à aider l'hôpital public à dépasser ce moment de décrochage qui nous inquiète tous légitimement. féliciter la ministre des solidarités et de la santé et dire que le travail engagé avec les fédérations et les nombreux interlocuteurs que nous avons consultés pour élaborer ce plan permet un bon plan, un vrai plan, un plan pour l'hôpital

acceptables, car elles sont insuffisantes. Je voudrais vous donner quelques pistes supplémentaires. Il faudrait que vous puissiez, dans le cadre d'un programme, donner leur autonomie aux hôpitaux, débureaucratiser l'hôpital, rendre le pouvoir à ceux qui soignent et, pourquoi pas, remettre en place des conseils d'administration plutôt que des conseils de surveillance, accepter de donner une juste rémunération aux personnels qui sont les moins bien payés en Europe et régionaliser l'organisation de la santé pour y impliquer les collectivités locales et se rapprocher des besoins de terrain. La

Ce 20 novembre marque le trentième anniversaire de la convention internationale des droits de l'enfant, que notre pays a signée le 26 janvier 1990, de même que 192 pays. Cependant, de nombreux droits de l'enfant peinent encore à être respectés. Je veux saluer tout particulièrement l'Unicef, qui oeuvre au quotidien pour le respect de cette convention dans le monde, convention qui introduit le concept d'intérêt supérieur de l'enfant et fait de ce dernier non plus un objet de droit, mais un sujet. saluer les bénévoles des centaines d'associations qui, partout sur nos territoires, s'investissent. Je veux enfin saluer les maires, qui jouent un rôle essentiel, particulièrement dans les Villes amies des enfants comme l'était ma ville de Bron, l'une des premières à adhérer à ce réseau lancé par l'Association des maires de France, dont le congrès se tient réalités. La France compte 1,8 million d'enfants et d'adolescents pauvres ; 17 % de ces enfants sont très jeunes, moins de 10 ans ; plus de 600 000 enfants vivent dans des conditions indignes et ce n'est pas le budget du logement que vous avez décidé d'amputer de près de 6 milliards d'euros sur le quinquennat qui améliorera la situation. Un enfant meurt tous les cinq jours de violence intrafamiliale ; 155 000 enfants sont victimes chaque année de violences sexuelles. Le récent rapport du Défenseur des droits relatif aux violences subies par les enfants au sein des institutions publiques souligne également qu'elles sont une réalité dans le quotidien des enfants et que le fonctionnement de ces institutions publiques est susceptible en lui-même d'induire des violences faites aux enfants dont elles ont la charge. Aussi, en ce jour anniversaire et alors que le Gouvernement vient d'annoncer un plan pour lutter contre les violences faites aux enfants, quelles décisions concrètes le Gouvernement compte-t-il prendre pour mieux protéger nos enfants ?

Vous le savez bien, madame la sénatrice, le Gouvernement n'a pas attendu ce trentième anniversaire ni même ma nomination à ce secrétariat d'État il y a désormais dix mois, pour oeuvrer en faveur des droits des enfants

l'action menée par Sophie Cluzel pour l'école inclusive ou encore le repérage précoce des enfants avec trouble du spectre de l'autisme, afin qu'ils soient mieux accompagnés, y concourent aussi. Je pense encore à la nécessité d'une justice adaptée, promue par la garde des sceaux, dans le cadre de la réforme de l'ordonnance de 1945. Pour autant, il est un droit sans lequel aucun autre droit n'est possible, c'est le droit à la sécurité, à la fois matérielle et affective. Le docteur Marie-Paule Martin-Blachais, dans le cadre d'une conférence de consensus, avait évoqué ce qu'elle appelait le « métabesoin ». C'est la raison pour laquelle, ce matin, le Président de la République a présenté à l'Unesco un certain nombre de mesures pour lutter contre les violences faites aux enfants. Vous avez rappelé un certain nombre de chiffres. Il est absolument inadmissible dans un pays comme le nôtre que les enfants puissent vivre ce type de violence. prévues pour garantir la sécurité de nos enfants partout, tout le temps, dans les institutions de la République- vous avez raison de le dire -, à l'école- je pense au cyberharcèlement -, mais aussi dans les institutions pour les enfants en situation de handicap ou encore dans les institutions de l'aide sociale à l'enfance. Il s'agit de garantir à tous les enfants qu'aucune grande personne en contact avec ces enfants ne puisse avoir été par le passé auteur d'actes pédocriminels. C'est l'une des mesures fortes de ce plan, madame la sénatrice.

Comme le revendiquent aujourd'hui 35 associations, ONG et collectifs, dont l'Unicef, il faut passer de la convention aux actes en s'engageant sur un objectif de zéro enfant dans la rue d'ici à 2022 et en créant un observatoire national de la non-scolarisation pour détecter les jeunes qui sont vulnérables.

M. le ministre Delevoye. Le Président de la République l'a toujours dit : pour qu'il y ait une réforme des retraites en 2025, il faut que le système soit équilibré. D'ailleurs, M. le Premier ministre l'a confirmé devant le Conseil économique, social indiquant que l'on ne pouvait pas laisser filer un déficit, que le fait de vivre avec un déficit n'était pas forcément le signe d'une bonne santé ou d'une bonne gestion, que, le rapport cotisants-pensionnés n'étant pas favorable, le système allait se dégrader. Il a même été précisé à Rodez que, si le déficit était entre 8 milliards et 10 milliards d'euros, il faudra dire

Monsieur le sénateur René-Paul Savary, je m'adresse à vous en tant que rapporteur pour l'assurance vieillesse, mais aussi en tant que membre du Conseil d'orientation des retraites. sociales, Alain Milon, et de son rapporteur général, Jean-Marie Vanlerenberghe, tous les travaux qui ont été engagés par le Sénat pour soutenir un système par points et toutes les contributions de la Haute Assemblée pour trouver un juste équilibre dans un système de répartition entre les jeunes actifs et les retraités. Il ne vous a pas échappé que le Conseil d'orientation des retraites tient son conseil d'administration demain et votre intervention s'inscrit probablement dans le droit-fil de celle que vous ferez devant les membres pluralistes de ce conseil pour justifier votre position et vos solutions,

L'engagement que nous avons pris avec un système par répartition, dont le plafond sera le plus élevé des pays développés, c'est d'assumer d'assumer l'universalité des droits, mais aussi la responsabilité qui consiste à ne pas faire porter sur les jeunes le poids d'un déficit que nous n'aurions pas réglé. Par conséquent, nous assumons, de la République, dans ceux du Premier ministre et dans les miens, que, à la suite de la remise de ce rapport, les décisions seront prises pour assurer aux futures générations un système juste, équilibré et solide, parce que nous ferons en sorte qu'il soit installé sur une base de zéro déficit.

mais ce pays est suffisamment chargé, soit on étudie des mesures d'âge, parce qu'avec une espérance de vie plus longue on peut peut-être songer à répartir un temps de travail plus long par rapport à un temps de retraite plus long. dans un système par points, vous introduisez un critère nouveau, qui est la valeur du point. Si le système n'est pas équilibré, plus le point est bas, plus les retraites sont basses et, au lieu d'avoir des gagnants et des perdants, vous pouvez n'avoir

la France rurale, parce que beaucoup de nos concitoyens y vivent, parce que l'on y trouve aussi des produits de grande qualité, solides- la gastronomie française est réputée -, mais aussi liquides.

dernier, la tolérance zéro concernant la consommation de boissons et la conduite. Nous avons déjà un arsenal répressif extrêmement fort.

vous avez raison : nos terroirs sont riches en gastronomie. Celui qui vous répond a soutenu pendant de longues années la Fédération nationale des bistrots de pays, le dernier commerce de proximité.

Nous sommes totalement mobilisés sur ce sujet. Il est vrai que, dans le cadre du comité interministériel de la sécurité routière du 9 janvier dernier, plusieurs mesures ont été proposées et mises en place pour lutter contre l'alcoolémie. Lutter contre l'alcoolémie ne signifie pas interdire de boire. Je vais être extrêmement clair, monsieur le sénateur : non, le Gouvernement n'envisage pas de revenir sur le taux d'alcool au volant et de l'abaisser à 0 gramme par litre de sang. Toutefois, monsieur le sénateur, chacun sait ici qu'il n'est pas sain de boire avant de prendre le volant. C'est cela que le ministre de l'agriculture a voulu rappeler. C'est une invitation à la citoyenneté, non seulement pour se protéger soi-même,

et peu efficaces, alors même que nous savons que nous avons besoin de les mobiliser pour la sécurité des Français. La n'ont pas d'autre choix que de prendre la voiture. Je suis totalement d'accord avec vous sur le fait qu'il faut consommer avec la plus grande modération. Cela ne doit pas nous empêcher

Il est important que l'on puisse aller déjeuner chez des amis ou chez des parents, sans avoir à craindre quoi que ce soit. Il est important que l'on puisse continuer à se déplacer. Nous vous remercions de veiller à ce qu'il en soit encore ainsi à l'avenir pour la liberté des ruraux

à Bercy, quand il le faut, on sait être pragmatique. À l'occasion de la fusion entre Fiat et le groupe PSA, l'État, actionnaire, a indiqué le chemin de l'efficacité en choisissant comme siège social Amsterdam.

aux Pays-Bas, ainsi que par la stabilité fiscale. L'État néerlandais utilise l'aéroport comme un point d'attraction pour les grandes entreprises internationales. Dans le même temps, le patron de Tesla, pour l'implantation de son usine en Europe, a choisi Berlin.

vous avez raison, les deux dossiers que vous évoquez, l'investissement dans une usine de batteries électriques, d'une part, ou l'investissement dans une usine de Tesla, d'autre part, montrent l'importance de mener une politique d'attractivité sur le territoire français. En termes d'attraction des projets

En 2018, Ernst & Young (EY) indiquait que la France accueillait plus de 330 projets d'investissements industriels, là où la Turquie, en deuxième position, en recevait environ 200 et l'Allemagne, que vous avez citée, 150. Donc factuellement, en 2018, la France accueille deux fois plus de projets industriels que l'Allemagne.

Il faut conclure ! ... la simplification est le dernier angle, et c'est celui dont nous nous emparons, notamment dans le cadre du pacte de production. La parole

Monsieur le ministre, lors du dernier comité État-régions, vous vous êtes prononcé contre une augmentation du transfert actuel de 7,5 % du premier pilier vers le second pilier de la PAC pour 2020, estimant que le taux actuel suffirait à garantir le bon financement des mesures jusqu'à la fin de la programmation. Or on sait que cette somme est bien insuffisante : les régions ont déjà consommé une grande partie, voire la quasi-totalité de l'enveloppe prévue pour les mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC) et les aides au bio. Ainsi, certaines restreignent déjà l'accès à ces financements, réservant par exemple les aides à la conversion en bio aux seuls projets portés par les jeunes agriculteurs. Comment comptez-vous répondre aux demandes communes des agriculteurs et des citoyens afin d'assurer les financements nécessaires à la transition agroécologique dans les territoires ?

aller au bout des aides qu'elles doivent apporter aux MAEC et au bio. C'est l'engagement qu'ont pris unanimement Régions de France et le Gouvernement, et je pense que c'est ce qui se produira en 2020,

en particulier dans la Drôme. J'associe donc mes deux collègues drômois Gilbert Bouchet et Bernard Buis à cette question. Dans la Drôme, 88 000 foyers ont été privés d'électricité et, hier soir, 7 000 étaient encore concernés. Pas d'électricité en cette saison, cela veut dire plus de chauffage, plus d'eau chaude, parfois même plus d'eau du tout, plus de communications possibles. Depuis six jours, cela a été ponctuellement dramatique et pourrait l'être encore si nous n'agissons pas. Cette situation est due à des chutes de neige abondantes précoces, avec une neige lourde et collante, à une période où les arbres portent encore leurs feuilles et sont donc plus sensibles au poids de la neige. Beaucoup sont tombés sur les routes et sur les installations électriques. Souvent aussi, les installations elles-mêmes ont cédé, pylônes compris. qui sont intervenus aussi vite qu'ils le pouvaient, mais surtout saluer le dévouement des maires et de nombreux élus qui sont restés sur le pont, nuit et jour, et tiennent bon, même même s'ils sont épuisés par cette épreuve. Aujourd'hui, cela fait six jours que cela dure et ils se sentent bien seuls face au désarroi et aux interrogations légitimes des habitants. Ce qui se passe au moment où je vous parle est grave. Les plus fragiles sont en danger et il faut y apporter des solutions sans tarder. À l'avenir, avec le changement climatique, ce type d'épisode neigeux risque de se reproduire. Aussi, madame la ministre, compte tenu de la situation et des dégâts très importants, je souhaite vous soumettre trois questions : que va faire l'État pour rétablir l'électricité tous les foyers encore concernés ? Quels nouveaux dispositifs pourraient être mis en oeuvre pour sécuriser les réseaux électriques afin d'éviter que cela ne se reproduise ? Peut-on envisager que ce type d'événement puisse être reconnu comme catastrophe naturelle ou trouver un autre moyen d'indemnisation ?

et je voudrais à mon tour rendre hommage aux élus, aux gendarmes, aux pompiers, aux renforts militaires, aux agents d'Enedis et de RTE, qui se sont mobilisés sans relâche. Vous l'avez dit, cet épisode Vous l'avez dit, cet épisode est dû à de la neige lourde, collante, tombée rapidement sur des arbres qui avaient encore des feuilles. De nombreux arbres sont tombés, qu'il a fallu déblayer

grêle. Nous n'avons donc pas besoin, dans ce cas particulier, de déclarer l'état de catastrophe naturelle. Ma question s'adresse à M. le ministre de l'action et des comptes publics. Monsieur le ministre, le Président de la République aime les élus- d'ailleurs, il n'a cessé de le répéter hier, lors du congrès des maires de France mais votre gouvernement a tout de même la fâcheuse habitude de s'immiscer dans les finances locales. Concernant la taxe d'habitation, François Baroin a eu raison de rappeler hier au Président de la République que vous aviez décidé de supprimer un impôt qui ne vous appartient pas. Il faut que la considération aille de pair avec le respect. De respect, il en est question quand votre gouvernement dépose sur le projet de loi de finances pour 2020 un amendement prévoyant qu'une partie des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) perçus par les départements franciliens et la Ville de Paris sera prélevée au profit de la Société du Grand Paris (SGP) ! Excusez du peu : 75 millions d'euros en 2020, puis 60 millions d'euros par an à partir de 2021 pour financer, tenez-vous bien, les engagements de l'État inscrits dans le contrat de plan État-région 2020-2022 sur les transports. Coût pour mon département : plus de 3 millions d'euros, alors même que l'Essonne pâtit d'infrastructures de transports surchargées et vieillissantes. Non content d'avoir reporté la construction de la ligne 18, qui devait dynamiser le plateau de Saclay, des Yvelines jusqu'en Essonne, ou le Charles-de-Gaulle Express, qui devait faciliter l'accès au village olympique en Seine-Saint-Denis, l'État nous ponctionne pour sa mauvaise gestion ! Je veux bien vous accorder que vous n'êtes pas les seuls responsables du passif de la SGP, mais quand on exerce des compétences, il faut en assumer les responsabilités et le financement. Aussi, ma question est simple, monsieur le ministre : quand le Gouvernement va-t-il cesser de dévitaliser les collectivités locales, et en particulier nos départements, au mépris des élus et des populations que nous servons ? Et cela, vous l'avez compris, n'est pas qu'un problème francilien

; l'autre vise effectivement à affecter une fraction des DMTO des départements de la petite couronne au financement de ces infrastructures. Cela répond à un besoin d'infrastructures, vous l'avez noté, mais vous auriez pu également relativiser le coût pour les départements, en rappelant combien les DMTO ont été dynamiques au cours des dernières années, ce qui relativise grandement la « ponction » évoquée, puisque vous avez utilisé ce terme. Au-delà, vous nous demandez comment le Gouvernement entend continuer à aider les collectivités territoriales et vous nous dites même craindre une forme de dévitalisation. Je vous répondrai en trois chiffres. Le premier concerne les dotations de fonctionnement. Le Gouvernement a fait le choix de la stabilité, et vous aurez l'occasion de constater dans le projet de loi de finances que le total des concours financiers de l'État aux collectivités passera de 48,3 à 49,1 milliards d'euros en 2020. Après 11 milliards d'euros de baisse de 2014 à 2017, il est juste et utile de rappeler cette stabilité. Le deuxième chiffre concerne le maintien des dotations d'investissement.

lui. Peut-être faudra-t-il un jour réfléchir à un gel total de tous les cofinancements dans nos territoires respectifs, pour mettre l'État face à ses responsabilités ? À mesure unilatérale, réponse unilatérale !

demande le retrait de l'ordre du jour de son espace réservé du jeudi 21 novembre au matin de la proposition de loi permettant à tout médaillé militaire ayant fait l'objet d'une citation à l'ordre de l'armée de bénéficier d'une draperie tricolore sur son cercueil. Acte est donné de cette demande. C'est raisonnable ! J'informe le Sénat que des candidatures pour siéger au sein de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à agir contre les violences au sein de la famille ont été publiées.

la convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) a suscité l'espoir de réelles avancées en faveur des enfants dans le monde, en développant leurs droits civils, économiques, politiques, sociaux et culturels. Cependant, trente ans après, le constat reste très préoccupant. Dans le monde, la misère et la pauvreté ne cessent de s'étendre, sans oublier les conflits armés, qui aggravent encore plus des situations déjà catastrophiques. En France, à une autre échelle, les droits des enfants ne sont toujours pas respectés. Quelque 3 millions d'enfants vivent dans notre pays sous le seuil de pauvreté. Les inégalités en matière de santé, de logement, d'accès à l'éducation ou aux loisirs demeurent. De larges débats doivent être menés sur ces problématiques et aboutir à des solutions concrètes. Pour la santé et le logement, je pense en particulier à l'outre-mer. et infantile (PMI) est criante, tout autant que la lutte contre les logements insalubres, les bidonvilles, qui pourtant devrait permettre d'assurer à chaque enfant des conditions de vie acceptables et dignes. Enfin, de manière générale, les enfants ne sont pas exempts en France d'agressions physiques ou morales, comme le harcèlement, la maltraitance, la pédophilie, l'exploitation sexuelle, dans dans un cadre familial bien souvent, mais aussi, et de plus en plus, dans un cadre scolaire ou médico-social. Je voudrais m'attarder un peu sur cette question des violences faites aux enfants. Les progrès sont évidents, notamment l'abolition récente des châtiments corporels, votée par le Parlement en 2018. Cependant, le dernier rapport de l'inspection générale des affaires sociales sur le sujet dévoilait en avril des chiffres terrifiants

Toutes les améliorations encore possibles ont été renvoyées aux conclusions du Grenelle sur les violences faites aux femmes L'amendement déposé par mon groupe visant à retirer le droit de visite et l'autorité parentale aux conjoints violents n'a pas été discuté. C'est accablant, car un conjoint violent est bien souvent un mauvais père, voire un père violent. Mais les violences faites aux enfants existent aussi dans la sphère publique. En témoigne le rapport annuel du Défenseur des droits, rendu public ce lundi 18 novembre, qui relève les violences ignorées ou banalisées au sein des institutions publiques. Il constate de fait un décalage entre les droits proclamés et les droits réels. Aussi, pour réduire cet écart, le même rapport formule vingt-deux recommandations, la première étant de conduire un état des lieux de ces violences institutionnelles afin de quantifier le phénomène et d'orienter les politiques publiques, état des lieux qui pourrait être mené par les délégations parlementaires aux droits des enfants que nous vous proposons de créer. Hélas ! le sort réservé à notre proposition de loi

et soucieuse de préserver une organisation efficace du travail parlementaire, la commission des lois a considéré que la création d'une huitième délégation n'était pas justifiée.

En outre, le travail des délégations pourrait s'appuyer sur les recommandations du Défenseur des droits, qui, rappelons-le, n'a aucun pouvoir législatif.

revanche, le Comité des droits de l'enfant de l'ONU préconisait dans ses dernières observations sur les rapports de notre pays en 2016 de « mettre en place une commission spécialisée dans les droits de l'enfant au Parlement ». Les deux positions sont donc bien différentes. Nous avons besoin au Parlement d'un véritable cadre de travail permettant une veille précise sur les droits des enfants et un contrôle de l'action du Gouvernement- c'est notre rôle de parlementaires -, notamment dans l'application de la convention. Mes chers collègues, ce trentième anniversaire de la CIDE ne doit pas être qu'une célébration. Il faut lui donner le sens d'un nouvel élan pour les droits des enfants. Avec l'inscription de ce texte à l'ordre du jour, dont je me félicite,

L'adoption, ce 20 novembre 2019, de cette proposition de loi transpartisane permettrait d'avancer en ce sens. Il est tout à fait possible de prendre une telle décision.

des enfants aux écrans, une proposition de loi, rapportée par Stéphane Piednoir, relative à l'interdiction de l'usage du téléphone dans les écoles et dans les collèges, ainsi qu'une proposition de loi relative à la suppression de la publicité commerciale dans les programmes jeunesse, sur l'initiative de M. Gattolin.

23.2 demande aux États de reconnaître le droit des enfants handicapés de bénéficier de soins spéciaux. Nous avons voté voilà quelques jours la proposition de loi visant à améliorer l'accès à la prestation de compensation du handicap, déposée par Alain Milon et plusieurs de ses collègues.

Oui, le contrat social est incomplet ! Certains de ses membres, les plus fragiles, ont été oubliés : ceux pour lesquels on évoque l'existence d'un « intérêt supérieur », mais qui semblent comme exclus de l'intérêt général. général. Les jeunes enfants ne manifestent pas. Ils ne votent pas. Et leur détresse est le plus souvent vécue à l'écart, dans la solitude. Le combat pour mettre l'enfant au coeur des actions publiques est engagé depuis des années. Il est mené sur toutes les travées de cet hémicycle, mais il n'est pas encore gagné. Pendant longtemps, la notion de droit des enfants n'existait pas. Ceux-ci étaient considérés non pas comme des sujets de droit, mais comme des individus sans statut spécifique. Le 20 novembre 1989, les Nations unies ont adopté à l'unanimité pour la première fois la convention internationale des droits de l'enfant, faisant ainsi écho aux mots prononcés à Genève en 1924, quand la Société des Nations adopta le premier texte international reconnaissant aux enfants des droits spécifiques et précisant les responsabilités des adultes : « [ ...] l'humanité doit donner à l'enfant ce qu'elle a de meilleur. C'est grâce à une sénatrice communiste, Marie-Claude Beaudeau, que le 20 novembre devint la Journée nationale des droits de l'enfant en 1996.

la proposition de loi de la députée Maud Petit contre les violences éducatives ordinaires, soutenue au Sénat notamment par Laurence Rossignol, ou la proposition de loi de Florent Boudié sur la rétention administrative des mineurs.

sur les enfants, à la réforme de l'ordonnance de 1945 de la garde des sceaux, à l'école à 3 ans du ministre Jean-Michel Blanquer, à la prévention et à la lutte contre la pauvreté, Cependant, nous ne pourrons dire que notre pays progresse tant que nous n'aurons pas réussi à éradiquer les violences faites aux enfants et à faire respecter leurs droits. Cette conviction, je sais que nous la partageons tous. Et c'est parce que nous la partageons que nous sommes en train de donner à l'enfant la place qui lui revient dans le contrat social, au coeur du contrat social. Depuis quelques jours, voire quelques semaines, associations, citoyens, élus organisent et célèbrent la convention internationale des droits de l'enfant. Ce matin, à l'Unesco, le Président de la République a pris des engagements forts, qui seront défendus par l'ensemble du Gouvernement. Jamais, dans l'histoire de notre pays, la conscience de l'enjeu et de l'urgence n'a été aussi aiguë. Ce matin également, un plan d'actions de lutte contre toute forme de violence était dévoilé par le secrétaire d'État Adrien Taquet. Oui, l'urgence- c'est notre responsabilité -est de protéger toujours plus, de détecter et d'alerter, pour que plus aucun espace ne soit laissé aux violences dont les enfants sont victimes Avec Adrien Taquet, secrétaire d'État chargé de l'enfance, et avec tous les membres du Gouvernement, nous avons la conviction qu'une société qui ne sait pas protéger et faire grandir ses enfants dans un monde apaisé et rassurant est une société qui transige avec ses valeurs les plus fondamentales. Et je sais pouvoir compter sur vous, au sein de vos commissions et de vos groupes de travail ! L'enjeu est que chacune et chacun se saisisse du sujet et agisse au quotidien, quel que soit son rôle dans la société.

La délégation aux droits des femmes, qui a été largement évoquée, est aussi très vigilante face aux discriminations qui peuvent intervenir dès l'enfance. Vous le savez, la convention internationale des droits de l'enfant a son propre comité de suivi, devant lequel notre pays fait régulièrement le point. La France a institué un défenseur des enfants,

des fonctions propres aux autorités administratives indépendantes. Il ne me semble effectivement pas utile d'ajouter une nouvelle commission, fût-elle parlementaire. Sur le fond,

à l'enfance en général. Je souhaite qu'il y ait un suivi globalisé des dépenses et des politiques engagées en matière de protection de l'enfance, soit par l'État, soit par les organismes sociaux ou familiaux, soit par les collectivités locales.

Sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales ni des commissions chargées des affaires européennes, les délégations parlementaires aux droits des enfants ont pour mission d'informer les assemblées de la politique suivie par le Gouvernement

L'article 3 de la convention insiste sur l'intérêt supérieur de l'enfant, qui doit être une considération primordiale. Dans des observations de 2013, le Comité des droits de l'enfant indiquait : « Ce n'est pas une obligation discrétionnaire

Au paragraphe 7, « le Comité note avec préoccupation que seul un nombre très limité de dispositions de la Convention sont reconnues comme étant directement applicables et que les principes et droits qui y sont consacrés ne sont pas dûment intégrés dans la législation nationale nationale ». Au paragraphe 9, « le Comité note avec préoccupation que les progrès réalisés en ce qui concerne l'élaboration d'une politique globale durable de mise en oeuvre de tous les droits consacrés par la Convention sont insuffisants et que les différentes stratégies relatives à l'enfance mises en oeuvre dans l'État partie ne contiennent pas d'objectifs mesurables ». Au paragraphe 12, « le Comité recommande à l'État partie de veiller à ce que le mécanisme de coordination soit doté d'un mandat clair et de pouvoirs et de ressources suffisants

le Comité note avec préoccupation que le Défenseur des enfants ne dispose pas de suffisamment de ressources et manque de visibilité au sein de l'institution du Défenseur des droits ». Je rappelle que, lorsqu'il a été créé, le Défenseur des enfants était indépendant. Ce n'est qu'en 2012 qu'il a été rattaché au Défenseur des droits.

du Conseil national de la protection de l'enfance. Exactement ! Ce conseil indépendant est susceptible de contrôler un peu et d'émettre quelques observations sur la mise en oeuvre de l'action gouvernementale.

Cette affirmation de Jean-Jacques Rousseau dans son essai sur l'éducation a certainement inspiré l'évolution constante des droits de l'enfant à travers les décennies. Nous avons en effet assisté à une meilleure prise en considération de la fragilité des enfants et, ainsi, à un renforcement de leur protection. Cette reconnaissance de droits spécifiques à l'enfant s'inscrit dans la lignée de l'affirmation des droits de l'homme, dont notre pays peut s'enorgueillir Depuis la ratification de la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, la France s'est engagée à faire primer les intérêts des enfants sur des intérêts concurrents. Je remercie par ailleurs le groupe CRCE d'avoir sensibilisé notre assemblée sur cette question avec cette proposition de loi que nous examinons le jour de l'anniversaire de cette convention, qui est aussi, depuis 1996- là encore, sur l'initiative du groupe communiste la Journée nationale de protection des droits de l'enfant. Cette protection a connu un tournant avec la loi du 6 mars 2000, qui a créé une nouvelle autorité administrative indépendante, le Défenseur des enfants, chargée de promouvoir et de défendre leurs droits. Le Défenseur des enfants a ensuite été rattaché au Défenseur des droits par la loi du 1 mai 2011 et incarné par l'un de ses adjoints, qui pilote le collège chargé de la défense et de la promotion des droits de l'enfant. Par ailleurs, au cours des dernières années, les initiatives législatives spécifiques se sont multipliées, avec de grandes lois générales sur la protection de l'enfance, comme la loi du 5 mars 2007 ou celle du 14 mars 2016, mais aussi avec des lois plus ponctuelles, comme la loi de lutte contre les violences éducatives ordinaires ou celle contre l'inceste. Cependant, comme le soulignent les rapports annuels du Défenseur des enfants, la protection des mineurs reste malheureusement perfectible en France. Les principales préoccupations concernent notamment les enfants immigrés et enfants de demandeurs d'asile, les « mineurs délaissés » pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, mais non adoptables, ainsi que la question des mineurs délinquants. Je souhaiterais également appeler votre attention sur une tribune publiée aujourd'hui par le directeur de l'association Aide et Action France-Europe, dans laquelle il sensibilise les pouvoirs publics sur le droit à l'instruction. Dans l'Hexagone, alors que ce droit est reconnu par la loi française pour tous les enfants, français et étrangers, âgés de 3 à 16 ans, près de 100 000 enfants, dont une majorité vit en squat, bidonville, dans la rue ou souffre d'un handicap, ne sont toujours pas scolarisés. Ces chiffres sont indignes de notre pays Par ailleurs, je regrette vivement que la proposition de loi contre les violences familiales que nous avons adoptée il y a quelques jours ait complètement occulté le problème des violences faites aux enfants et que tous nos amendements sur le sujet aient été rejetés.

J'envisage également avec mon groupe de déposer une proposition de loi visant à favoriser l'adoption simple des mineurs délaissés. Nous examinons donc aujourd'hui la proposition de loi du groupe CRCE visant à créer une nouvelle délégation parlementaire consacrée aux droits des enfants. Si nous comprenons et partageons l'intention louable qui sous-tend cette proposition de loi, nous considérons néanmoins que la multiplication des délégations, ou encore des organismes extérieurs aux assemblées, éparpille le travail parlementaire, lui faisant nettement perdre en efficacité. existe déjà cinq délégations sénatoriales, dont l'efficacité est parfois questionnée. Ainsi, les propositions de ces délégations ne sont pas systématiquement suivies en commission, et elles disposent de moyens de fonctionnement moins importants que les commissions permanentes, limitant considérablement leur pouvoir d'initiative. Notre groupe est particulièrement attaché au débat et au travail parlementaire, tant législatif que de contrôle. Les initiatives de groupes de travail transpartisans, voire entre les deux assemblées favorisent les échanges et le consensus. Malheureusement, l'expérience montre que leurs travaux n'aboutissent pas à des textes concrets votés par l'ensemble des parlementaires. C'est la raison pour laquelle la grande majorité de notre groupe votera contre cette proposition de loi- non pas contre la nécessité de faire de la protection des droits de l'enfant une priorité, mais contre la création d'une délégation dont l'efficacité ne sera certainement pas au rendez-vous. Nous considérons que, pour améliorer concrètement la situation des enfants victimes de violences ou d'injustices sociales, la voie législative est indispensable. La parole

la discussion de la proposition de loi présentée par nos collègues du groupe CRCE est l'occasion de dresser un bilan de l'application de la convention internationale des droits de l'enfant, la CIDE, dont nous fêtons aujourd'hui même le trentième anniversaire de la signature. Ce texte révolutionnaire

cette convention. Parmi ces réformes figurent notamment la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance ainsi que celle du 10 juillet 2019- donc, très récente -relative à l'interdiction des violences éducatives ordinaires. Je rappelle que l'adoption de cette dernière loi a permis à la France de se conformer aux exigences énoncées à l'article 19 de la convention.

à l'Unesco, l'objectif de donner à tous les enfants les mêmes chances de départ dans la vie. Des mesures ambitieuses ont déjà été prises : renforcement de l'accès des enfants issus de familles pauvres aux crèches amélioration de l'accueil des élèves en situation de handicap ; création du dispositif des petits-déjeuners à l'école- qui n'est pas sans nous rappeler Mendès France aide à la mise en place d'une tarification sociale des cantines ; division par deux du nombre d'enfants par classe dans les écoles de quartiers défavorisés ; obligation d'instruction des enfants dès l'âge de 3 ans. Il s'agit là de six mesures importantes en matière de politique de l'enfance.

pour répondre aux besoins des enfants qui grandissent dans la pauvreté et l'exclusion. En France, 2,8 millions d'enfants vivaient sous le seuil de pauvreté en 2017, soit un enfant sur cinq. C'est non seulement non seulement considérable, mais intolérable ! Par ailleurs, d'importants efforts sont encore nécessaires pour venir à bout de toutes les formes de violence à l'égard des enfants, pour mettre fin au travail infantile, éradiquer le phénomène du tourisme sexuel impliquant des enfants, renforcer la protection des enfants migrants, à commencer par les mineurs non accompagnés, améliorer le sort des enfants atteints d'un handicap. Outre la mise en place de ces nombreuses mesures, nous devons réfléchir à la possibilité d'accorder de nouveaux droits aux enfants. En 2014, un groupe de travail présidé par l'ancien président du tribunal pour enfants de Bobigny, Jean-Pierre Rosenczveig, qui est une autorité non seulement judiciaire, mais aussi morale par son expérience en ce domaine, avait formulé pas moins de 120 propositions, dont l'abaissement à 16 ans de l'âge du droit de vote. La création de délégations parlementaires aux droits des enfants figurait également parmi les propositions de M. Rosenczveig. En 2003, l'Assemblée nationale a adopté une proposition de loi allant dans ce sens. Toutefois, ce texte n'a jamais été inscrit à l'ordre du jour de notre assemblée. C'est la raison pour laquelle, j'imagine, le groupe CRCE a déposé la proposition de loi soumise aujourd'hui Ce texte part d'une bonne intention. Cependant, notre groupe n'y est pas favorable. La problématique des droits de l'enfant est certes transversale, mais nous craignons que des délégations qui y seraient spécifiquement dédiées n'empiètent sur le périmètre des commissions permanentes, à commencer par celles des lois et des affaires sociales. revanche, nous serions tout à fait ouverts à ce que soit instauré un débat annuel devant le Parlement sur les politiques d'aide à l'enfance. l'enfance. Nous considérons que chaque chambre doit conserver sa liberté de dessiner l'architecture de ses organes d'évaluation et de contrôle. C'est une question qui revient de façon assez régulière, mais la création de nouvelles délégations nécessiterait sans doute une concertation préalable entre les deux assemblées dans la mesure où la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale date maintenant de plus de seize ans. Par ailleurs, nous constatons avec satisfaction que le contrôle du respect des droits de l'enfant occupe déjà une place importante dans les travaux du Sénat. Pour s'en convaincre, il suffit d'énumérer les rapports d'information

Il convient aussi de rappeler que la commission des lois auditionne régulièrement le Défenseur des droits, qui est notamment chargé de la défense et de la promotion des droits de l'enfant, avec la Défenseure des enfants. J'ajoute que la commission des affaires européennes est également compétente pour traiter des questions relatives aux droits de l'enfant. Je viens moi-même de la saisir d'une proposition de résolution européenne sur la protection des enfants franco-japonais, en parallèle d'une proposition identique identique en droit purement français. Enfin, notre assemblée sera prochainement amenée à se pencher sur la réforme de la justice pénale des mineurs. D'autres sujets mériteraient sans doute un examen approfondi. Je pense notamment au placement en rétention administrative des mineurs étrangers ainsi qu'à la transcription sur l'état civil français des enfants nés d'une GPA à l'étranger, que nous retrouverons sans doute dans le débat sur le projet de loi Bioéthique. Nos travaux doivent, de préférence, s'inscrire dans le cadre des commissions permanentes, des missions d'information et des commissions d'enquête. Nous savons tous quelles difficultés nous rencontrons, le mercredi et le jeudi, à courir d'une commission ou d'une délégation à l'autre, ratant une partie des débats. Pour toutes ces raisons, le groupe La République En Marche votera contre la présente proposition

ans après l'adoption de la convention internationale des droits de l'enfant, force est d'observer que, malgré des avancées réelles, le constat reste encore très préoccupant. Ma collègue Christine Prunaud a répondu aux arguments bien faibles, pour ne pas dire étranges de Mme la rapporteure pour expliquer le rejet de notre proposition de loi. Mais permettez-moi d'y revenir. Je dois vous dire que ces raisons, purement formelles, me sidèrent. Comment peut-on oser opposer à une problématique aussi importante que celle des droits des enfants des questions d'optimisation et d'efficacité ? Toute initiative qui permet la prise en compte et la promotion des droits des enfants et de l'égalité devrait constituer une avancée, d'autant que la création de ces délégations est également une recommandation du Comité des droits de l'enfant de l'ONU. Comment nier que, au même titre que la délégation aux droits des femmes, cette délégation aux droits des enfants a toute sa place et sa légitimité au sein de la Haute Assemblée La question des violences faites aux enfants, par exemple, a été développée par ma collègue. Cette délégation aux droits des enfants pourrait se saisir pleinement du sujet en étant à l'initiative de recommandations de rapports visant à aiguillonner le travail du Gouvernement et éclairer notre société sur les réalités des situations et, surtout, sur le chemin qui reste à parcourir pour considérer les enfants comme de vrais sujets de droit. Elle pourrait même, de sa propre initiative, déposer des amendements dans les différents projets de loi. Un autre champ d'action à investir pourrait être l'harmonisation de l'accueil des enfants dans les services d'aide sociale à l'enfance, laquelle est placée sous l'autorité des conseils départementaux, aux moyens disparates sur notre territoire, et dont dépend l'accueil des mineurs non accompagnés, autrement dit des mineurs isolés étrangers dont la situation se révèle de plus en plus inquiétante ; ces mêmes mineurs- des enfants donc ! -qui se retrouvent parfois privés de liberté dans les centres de rétention administrative. Ce dernier sujet parfaitement la transversalité des problématiques à traiter en matière de droits des enfants, qui relèvent à la fois, s'agissant de l'enfermement des enfants, par exemple, des compétences de la commission des affaires sociales et de la commission des lois.

Comme nous l'indiquons dans l'exposé des motifs de notre proposition de loi, d'après les derniers chiffres de la Banque mondiale, d'ici à 2050, 140 millions de personnes pourraient être amenées à migrer en raison de l'aggravation des effets du changement climatique. Parmi elles, bien évidemment, de nombreux enfants, aussi vulnérables face à ces changements climatiques que face à la pollution atmosphérique. Comme l'a récemment révélé l'OMS, la pollution de l'air a tué 600 000 enfants de moins de 15 ans en 2016 dans le monde et affecte plus de 90 % des enfants de la planète. Dans ce cadre, le 23 septembre dernier, seize enfants du monde entier ont déposé plainte auprès du Comité des droits de l'enfant des Nations unies. Ces jeunes militants ont attaqué cinq pays pollueurs, dont la France, pour protester contre le manque d'engagement des gouvernements face à la crise climatique et demander aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour protéger les enfants des effets dévastateurs du changement climatique. Au lieu de pointer du doigt cette action, la France et son parlement s'honoreraient à travailler sur le sujet en entendant, pour une fois, la voix d'enfants qui se saisissent eux-mêmes de leur droit à vivre sur une planète plus saine et à respirer un air moins pollué. Quelle Quelle commission permanente pourrait s'emparer d'un sujet aussi complexe ? La délégation aux droits des femmes, me répondrez-vous peut-être.

le droit d'allaiter pendant le temps de travail reconnu aux femmes fonctionnaires », qui résulte d'un amendement introduit par la délégation au droit des femmes dans la loi de transformation de la fonction publique. Comme le disent les jeunes : j'hallucine

enfants, qui n'est pas qu'une date symbolique, tâchons de nous en souvenir ! Toute la société, au premier rang de laquelle les législatrices et législateurs que nous sommes, a le devoir et la responsabilité de donner aux enfants les moyens de construire leur avenir, un avenir fondé sur des valeurs de progrès, de solidarité, de fraternité, de paix, bannissant la violence, quelle que soit la forme qu'elle puisse revêtir. Pour cela, il nous appartient de faire acte de vigilance, de proposer et d'être à l'initiative de nouveaux droits effectifs pour les enfants. C'est le rôle du Parlement, et c'est le sens de notre initiative aujourd'hui.

Il apparaît évident que l'humanité ne pourra se prévaloir d'avoir fait progresser les droits de l'homme tant qu'elle n'aura pas réussi à éradiquer le fléau des violences faites aux enfants et tant qu'elle ne sera pas parvenue à faire respecter leurs droits fondamentaux. Cette volonté est universelle. Elle est aussi celle de notre pays, celle des pouvoirs publics, de la représentation nationale ainsi que de la société civile. Cette volonté commune, nous la partageons tous, et elle nous engage tous. Elle nous engage à agir. Elle nous engage à être efficaces pour faire respecter ces droits. Elle nous engage à nous occuper de l'enfance meurtrie, mutilée, de cette enfance qui souffre et subit parfois dans le silence. En ce jour du trentième anniversaire de la convention internationale des droits de l'enfant, la proposition de loi tendant à la création de délégations parlementaires aux droits des enfants permet de rappeler que la protection de l'enfant et son intérêt supérieur doivent être une préoccupation constante du législateur, comme du Gouvernement. À cet égard, cette initiative de notre collègue Éliane Assassi mérite d'être saluée. Dans le cadre de ses structures internes actuelles, le Sénat se saisit régulièrement de ces sujets et peut veiller avec efficacité au respect des droits des enfants. Aussi, au regard du travail effectué par les instances actuelles et des moyens à la disposition des parlementaires pour contrôler l'action du Gouvernement, la création d'une nouvelle délégation spécialisée ne semble pas justifiée. En premier lieu, les commissions permanentes mènent régulièrement, dans leurs champs de compétences respectifs, des travaux législatifs ou de contrôle sur la situation des enfants. Sont les plus concernées : la commission des affaires sociales, dans le cadre de ses compétences en matière de santé, de politique familiale, d'aide et d'action sociales la commission de la culture, sur les sujets relatifs à l'enseignement scolaire et à la jeunesse ; la commission des lois, s'agissant notamment des mineurs délinquants et des évolutions de l'ordonnance du 2 février 1945. En deuxième lieu, des missions ou des missions communes d'information sont également créées pour examiner des politiques publiques en faveur des enfants, comme en 2019 sur les politiques publiques de prévention, de détection, d'organisation des signalements et de répression des infractions sexuelles susceptibles d'être commises par des personnes en contact avec des mineurs dans le cadre de l'exercice de leur métier ou de leurs fonctions. En troisième lieu, la délégation aux droits des femmes travaille de manière plus spécifique sur la situation des enfants à l'occasion de travaux consacrés à la situation des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. En dernier lieu, le Sénat mène des travaux relatifs aux droits de l'enfant dans un cadre plus large que les commissions permanentes et les délégations. C'est le cas à travers la participation des sénateurs aux assemblées parlementaires ou encore à l'occasion des questions au Gouvernement. Il existe ainsi une palette de moyens mis à la disposition des parlementaires en ce qui concerne le respect des droits des enfants. Aussi, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, la création d'une nouvelle délégation pour mettre en place une veille et un contrôle plus assidus du respect des droits des enfants ne semble pas opportune. Par ailleurs, il convient de préserver l'efficacité du travail parlementaire accompli par les structures déjà existantes. Multiplier des organismes conduirait à un alourdissement inutile. Aussi,

Madame la présidente, mes chers collègues, en ce trentième anniversaire de la convention internationale des droits de l'enfant, je tiens à dire que je soutiens la proposition de loi qui est présentée par le groupe CRCE.

cette proposition de loi pour pouvoir mieux défendre les droits des enfants.

de la France qu'elle mène ce combat. Ce serait l'honneur du Parlement de voter cette proposition de loi, et je regrette profondément que le poids administratif ne le permette pas.

« rien n'est plus important que de bâtir un monde dans lequel tous nos enfants auront la possibilité de réaliser pleinement leur potentiel et de grandir en bonne santé, dans la paix et dans la dignité ». Ces mots de Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations unies, trouvent, je crois, un écho en chacun de nous. Comme citoyen, comme parent, comme sénateur, nous avons tous à coeur de défendre l'intérêt supérieur de l'enfant et de conforter l'enfant comme sujet de droit. C'est ce sentiment plein d'humanité, que je partage évidemment, qui a animé les auteurs de cette proposition de loi. Ainsi, comme son titre l'indique, ce texte a pour objectif de constituer une délégation parlementaire aux droits des enfants. Pour cela, l'article unique institue tout d'abord dans chaque assemblée une délégation parlementaire aux droits des enfants de trente-six membres, choisis à la représentation proportionnelle des groupes. ensuite ces délégations d'assurer le suivi de la politique des droits des enfants et leur permet d'être saisies de projets ou de propositions de loi, sur demande du bureau, d'un président de groupe, d'une commission ou sur sa propre initiative. Il prévoit enfin la remise d'un rapport d'activité annuel, comprenant le cas échéant des « propositions d'amélioration de la législation et de la réglementation » sur leur domaine de compétence. compétence. Dans un contexte d'inflation législative, que nous devons combattre, je suis convaincu que chaque texte qui est soumis au Parlement doit répondre à cette question essentielle et simple, qui fait fi des considérations partisanes : est-il réellement efficace compte tenu des objectifs fixés ? ? Malgré les bonnes intentions indéniables de ce texte, je crois que la réponse est négative, d'une part, au regard du cadre juridique existant et, d'autre part, quant au choix organique pour les atteindre. La protection des droits des enfants est un sujet d'importance encadré à la fois par le droit international et national. De multiples mécanismes de protection ont été retranscrits à la suite de l'adoption de la convention internationale des droits de l'enfant en 1989. Sur le plan intérieur, si de nombreux organismes de l'État, notamment le ministère des solidarités et de la santé, ainsi que les collectivités territoriales participent à la politique de l'enfance, la France dispose aussi de plusieurs instances se consacrant spécifiquement à la question, notamment le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, ou encore le Défenseur des droits. En outre, la France a jusque très récemment adopté un certain nombre de textes et de mesures destinés à mieux protéger les droits des enfants, comme la loi du 5 novembre 2015 tendant à clarifier la procédure de signalement de situations de maltraitance par les professionnels de santé, initiée

À ce titre, je ne suis d'ailleurs pas opposé, chère Joëlle Garriaud-Maylam, à une réorganisation de celles qui existent. Si la question de la création d'une délégation aux droits des enfants n'est pas nouvelle, je suis toutefois

Bien sûr, ce sujet touche des convictions profondes. Il est donc normal et souhaitable de pouvoir en débattre, y compris au sein de notre groupe, où la liberté de chacun est toujours garantie. C'est pourquoi j'entends parfaitement les arguments avancés par notre collègue Garriaud-Maylam, que je connais bien et dont je sais le travail et l'engagement depuis de nombreuses années sur ce qui, j'en conviens, doit être une préoccupation majeure. doit être une préoccupation majeure. Mais je crois profondément que notre arsenal juridique, sans doute encore imparfait, permet d'y répondre sans la création d'une délégation spécialement dédiée. Je suis tout aussi convaincu que les enfants, ces citoyens en devenir, doivent être des acteurs de leur propre avenir et, par là même, de leurs droits, à condition bien entendu de les connaître. Cela passe, mes chers collègues, encore et toujours, par l'éducation des parents et par une école de la République qui instruit.

En ce jour, choisi par le Parlement en 1996 pour être la Journée mondiale de défense et de promotion des droits de l'enfant, il est nécessaire de rappeler que protéger les plus jeunes est indispensable. Il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l'enfance. En France, 19 000 enfants sont maltraités, 76 000 sont en danger dans un contexte familial dégradé, 240 000 sont placés ou pris en charge et 150 000 quittent chaque année le système scolaire. La France n'est pas assez riche d'enfants pour qu'elle ait le droit de négliger tout ce qui peut en faire des êtres sains. Analyser les failles du droit sur le sujet participe de leur protection. À ce titre, je salue la volonté de nos collègues, dont la justesse dans l'idée ne fait pas de doute. C'est dans l'application que j'émets en revanche quelques réserves.

que nous traitons aujourd'hui. Au niveau de la méthode, ces propositions de loi tendent à introduire un article dans l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Or la multiplication excessive des structures internes au Parlement rend la lecture de son fonctionnement complexe pour le citoyen et contribue à la mise en danger du modèle de représentation démocratique, déjà menacé par une défiance sans précédent à l'égard du politique. Le président de la commission des lois de l'époque, Pascal Clément, avait exprimé des réserves à l'égard de la création de nombreuses délégations, qui lui paraissait constituer une manière de contourner la limitation à six du nombre des commissions permanentes. Je pense qu'il serait plus opportun de redéployer les compétences actuellement dévolues aux commissions permanentes et délégations existantes, ou de faire appel aux outils que sont les commissions d'enquête et missions d'information, plutôt que d'épaissir le millefeuille. La France peut mieux faire, comme l'indique le Conseil français des associations pour les droits de l'enfant. Notre rôle, c'est d'agir par le droit, sur le droit ! Or créer une instance non normative sur un sujet aussi crucial peut envoyer un signal très flou à la société civile, créant une forte attente sur le sujet ; attente qui sera forcément déçue, puisqu'une délégation nourrit, mais ne fait pas la loi En effet, une délégation, ce sont des administrateurs qui rédigent des synthèses, des rapports, ce sont des auditions, des visites, des réunions, beaucoup de travail de fond, mais ce n'est pas la production d'actions. Et des outils, il en existe déjà beaucoup Pour nos enfants, il y a d'abord des principes fondamentaux, rappelés dans le code civil et dans le code de l'action sociale et des familles. La convention internationale des droits de l'enfant de 1989 a créé un statut très protecteur, mais ne suggère en rien la création de délégations. Il y a ensuite des lois, celle du 10 juillet 1989 relative à la prévention des mauvais traitements, celle du 17 juin 1998 sur les infractions sexuelles, celle du 9 mars 2004 allongeant la prescription pour les délits commis sur des mineurs, celle du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance et, bien sûr, celle du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant. J'ajoute tous les travaux du Sénat, rappelés par notre collègue Muriel Jourda. Il Il y a enfin des institutions veillant à l'application de ces lois et principes : l'Unicef aux plans mondial et européen, l'Observatoire national de l'enfance en danger et, surtout, le Défenseur des droits pour appliquer la convention en France. femme et mère de famille, il est évident que je suis sensible à ce sujet des droits de l'enfant. Nous devons renforcer les moyens de les protéger, mais ce n'est, hélas, pas la mission d'une délégation. La discussion générale est close.

! Contrairement à ce que vous pensez, c'est pleinement en rapport avec le droit des enfants, cette recommandation émanant directement d'un rapport du Défenseur des droits et du Défenseur des enfants

Nous examinons cette proposition de loi dans un contexte particulier : aujourd'hui, nous fêtons le trentième anniversaire de la convention internationale des droits de l'enfant, adoptée à l'unanimité de l'assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989. Cette Journée internationale des droits de l'enfant intervient quelques jours après la discussion du rapport annuel du Défenseur des droits sur les violences institutionnelles que subissent les enfants dans notre pays. Les chiffres sont plus qu'alarmants 25 % des collégiens déclarent avoir été victimes d'atteintes en ligne, plus de 50 % des mineurs accueillis dans les foyers de l'enfance n'ont pas reçu de visite depuis trois mois, un enfant en situation de handicap, en particulier mental, est quatre fois plus exposé aux violences sexuelles que les autres enfants ... Je pourrai encore rappeler que 70 % des enfants issus de l'ASE sortent sans diplôme. Au-delà de l'émotion et de l'indignation que ce rapport suscite, il pointe une réalité à laquelle nous devons réagir. Je le rappelle, un viol a lieu toutes les heures et 73 000 enfants sont victimes de violences. Je partage la volonté de renforcer le contrôle exercé par le Parlement sur le respect des droits de l'enfant, comme nous pouvons exercer ce contrôle sur le droit des entreprises. C'est pourquoi je voterai cette proposition de loi et souhaite m'y engager pleinement. J'ai toujours pensé que la protection de l'enfance et le respect des droits de l'enfant dépassaient les clivages et les couleurs politiques. Très bien ! Voter la création d'une délégation aux droits de l'enfant constituerait un message fort envoyé au monde de la protection de l'enfance. Cela s'inscrirait également dans la continuité des annonces faites par le Président de la République et des vingt-deux mesures annoncées aujourd'hui par Adrien Taquet, qui permettront, nous le souhaitons, de lutter contre les violences faites à nos enfants.

rapport ! Je savais bien, à l'issue des travaux de la commission, que notre proposition de loi ne serait pas adoptée aujourd'hui, en particulier à la demande de la majorité sénatoriale.

la France ne fait pas assez d'efforts pour comprendre, prévenir et combattre les injustices et les violences que subissent les enfants. Est-il vraiment

à lutter contre la maltraitance et à la prévenir pour faire en sorte que nous n'ayons plus tous ces enfants qui souffrent en secret et en silence pendant des années avant d'être pris en charge et protégés.

c'est de faire en sorte que les enfants soient protégés. Bien sûr ! Le lien automatique que vous semblez faire entre une délégation sénatoriale aux droits de l'enfant et l'amélioration de la protection de l'enfance n'existe pas. Bravo ! Ce n'est pas cela ! Il existe d'autant moins

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, nous abordons, sur l'initiative de mon groupe, la question du maintien et du développement des auto-trains et des trains de nuit. Alors que l'accord de Paris doit s'appliquer dès 2020, il nous semble utile de revenir sur les outils concrets de respecter les engagements qu'elle a contractés pour elle-même. Notre pays peine à atteindre les objectifs de réduction de 27 % de ses émissions à l'horizon de 2028 par rapport à leur niveau de 2013 et de 75 % d'ici à 2050. Selon les bilans de l'Observatoire climat-énergie des ONG, les objectifs de la stratégie nationale bas-carbone n'ont pas été atteints depuis 2016. Les émissions de gaz à effet de serre ont dépassé, en 2017, de 6,7 % le budget que l'État s'était fixé. Le dépassement était de 4,5 % en 2018. Le secteur des transports, qui représente environ 30 % de ces émissions, a dépassé de 12,6 % son budget carbone en 2018. Cela, alors même que les objectifs de report modal sont à la traîne. Ainsi, le résultat de 2018 pour le report modal du transport de marchandises est en recul de 23 % sur l'objectif, avec seulement 10,9 % de parts de marché. On voit bien la tendance qui se dessine, c'est celle d'une politique nationale du tout-routier et du tout-aérien, reléguant le ferroviaire au rang de parent pauvre des politiques publiques.

il y a une réalité, celle d'une planète inhabitable et d'une humanité condamnée par l'augmentation des températures à un niveau supérieur à 2 degrés. Nous devons réagir ! Les marches pour le climat en France et dans le monde, l'action judiciaire engagée contre la France par une jeunesse outrée de tant d'inconséquence devraient nous faire réfléchir. La dernière tribune d'experts parue dans nous y exhorte, d'autant que les changements pourraient être plus rapides que prévu. Le Président Macron appelait au « », mais toutes mais toutes les politiques menées sont à contre-pied de ces objectifs, puisqu'elles cassent les services publics, qui sont pourtant des outils extraordinaires pour la transition écologique et, singulièrement, pour le service public ferroviaire. La SNCF, dont l'État est l'unique dont l'État est l'unique actionnaire, se perd ainsi depuis des décennies dans une stratégie du tout-TGV et de la rentabilité à tout prix, sacrifiant ses autres activités jugées trop peu rentables : le fret, l'auto-train et les Intercités. La logique de casse du service public est bien toujours la même : segmentation, externalisation et socialisation des pertes. On asphyxie le service public en le rendant inopérant et marginal pour l'abandonner ensuite ou le céder au privé au motif de sa dégradation et de son inadéquation avec la demande. Le fret a été dépecé, au gré des différents plans d'entreprise, le comble étant aujourd'hui le renoncement à la ligne Perpignan-Rungis. Une démonstration, s'il le fallait, que la concurrence ne peut être l'alpha et l'oméga des politiques, publiques puisque le marché ne reconnaît pas l'intérêt général, ne s'intéressant qu'au profit immédiat. Le marché ne pense pas le temps long, il est dans le rendement immédiat. Il est donc incapable de répondre aux enjeux écologiques de développement du fret ferroviaire. du fret ferroviaire. J'avais interpellé l'ancien président de la SNCF sur l'arrêt du service auto-train. Là encore, le scénario est le même. En trente ans, le service a perdu 80 % de trafic et les trains auto-couchettes ont totalement disparu, d'une politique coupable de rétraction de l'offre. Les possibilités de substitution promues par l'entreprise- le transport des voitures par camion ou leur acheminement par la route avec un chauffeur

pour permettre la reprise de cette activité prisée par certains publics, tels les seniors ou les motards. Enfin, sur la question particulière des trains Intercités, la situation est différente. En effet, l'État a ici, en tant qu'autorité organisatrice, une responsabilité particulière, par l'intérêt de ces lignes en termes d'aménagement du territoire. Alors qu'il existait plus de soixante lignes de trains Intercités au début des années 2000, les différents gouvernements, aidés par la SNCF, ont taillé dans l'offre. Aujourd'hui, il ne reste que six trains Intercités de jour et deux trains trains Intercités de nuit. Pourtant, l'offre continue d'être sabotée par les bugs informatiques constants, les travaux et les suppressions de dernière minute. constaté, en 2017, 47 % de déprogrammations sur le Paris-Irún. Le taux d'occupation de l'ordre de 47 % apparaît, dans ces conditions, un exploit, qui pourrait largement être dépassé. Mme Borne annonce comme un succès un investissement de 30 millions d'euros pour rénover le matériel, faute de le remplacer. Pourtant, les sommes accréditées dans le cadre du compte d'affectation spéciale sont en diminution de 47 millions d'euros. Comment comprendre Pis, nous craignons, au regard de la faiblesse des investissements, le non-remplacement des sièges inclinables, ce qui serait dramatique pour l'attractivité du train de nuit. Nous attendons sur cette question des engagements fermes de la part du Gouvernement. Notre groupe a déposé et fait adopter, dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités (LOM), un amendement engageant le Gouvernement à étudier le déploiement des trains de nuit. Cet amendement, voté ici, au Sénat, a été conservé à l'Assemblée nationale, ce qui signifie qu'il s'agit d'un objectif largement Les usagers sont eux aussi très attachés à ce service, comme en témoigne le succès de la pétition « Oui au train de nuit ! », qui a recueilli plus de 160 000 signatures. Cette pétition demande la mise en chantier de quinze lignes nationales de nuit et de quinze lignes internationales à l'horizon de 2030. Une perspective qui permettrait, selon les estimations de l'association à l'origine de la pétition, d'économiser l'émission de 1,5 million de tonnes de CO2. Les trains de nuit présentent de nombreux avantages. Ils sont peu énergivores ; l'avion émet quatorze à quarante fois plus de CO2 que le train. Ainsi, sur les 164 millions de passagers aériens, 86 millions pourraient, avec une offre à la hauteur, se reporter sur les trains de nuit. Ce mode de transport répond également aux enjeux de lutte contre la pollution aux particules fines, qui tue chaque année 48 000 personnes. Peu coûteux, ce « report modal » sur le réseau classique a l'avantage d'être beaucoup moins onéreux

Il constitue un outil utile d'aménagement du territoire, notamment grâce aux liaisons transversales et à la possibilité d'une desserte fine. Par son prix attractif, il permet de lutter contre les fractures sociales. Pourtant, aujourd'hui, les analyses « officielles » sur ce mode de transport lui sont largement défavorables. Elles sont partielles et partiales. Il est injuste de pointer spécifiquement le déficit de cette offre. Le déficit du train de nuit est de 18 euros par voyageur sur 100 le déficit Intercités de jour est de 23 euros, quand celui des TER avoisine les 30 euros. Et je ne vous parle même pas des gouffres financiers de certains projets de TGV Par ailleurs, ce manque de rentabilité est à relativiser : la route coûte elle aussi très cher et même plus cher ! Ainsi, les chercheurs de l'université technique de Dresde ont évalué récemment ces dépenses à 50,5 milliards d'euros pour la France. Toujours selon cette étude, le le coût des accidents de la route serait de 16,8 milliards d'euros en 2018. À cela, il faut ajouter des dépenses globales des administrations de 15,2 milliards d'euros par an, dont 12,9 milliards d'euros pour les collectivités je ne parle pas non plus de toutes les aides fiscales aux chargeurs routiers et autres exonérations de TICPE ! Quant à l'avion, celui-ci bénéficie d'un traitement de choix : subventionnement des aéroports régionaux et kérosène détaxé, ce qui représente pour le budget un coût de 3 milliards Le choix de l'abandon du rail sous toutes ses formes est donc un choix politique, celui du désengagement de l'État des secteurs clefs de l'économie au profit d'un système ubérisé et d'une économie libéralisée. Nous sommes aujourd'hui dans un marché des transports structuré non pas autour des besoins des usagers et des territoires, mais autour de politiques marketing fondées sur le développement des offres low cost et, donc, sur le dumping social et environnemental. Une situation qui, vous l'avouerez, porte des risques lourds pour la sécurité des usagers et des personnels. Nous appelons donc très directement le Gouvernement à changer de braquet. L'État doit prendre ses responsabilités. Premièrement, parce qu'il est l'actionnaire unique de la SNCF. sa qualité d'autorité organisatrice, d'affecter de nouvelles ressources à cette offre. Cela passe par un certain nombre de propositions sur lesquelles je n'ai pas le temps de m'étendre. Je pense que la France est confrontée à de nombreux

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je tiens à remercier nos collègues du groupe CRCE pour la tenue de ce débat sur le thème : « Pour répondre à l'urgence climatique par le développement ferroviaire : promouvons les auto-trains et les Intercités de nuit. nuit. » En tant que sénatrice des Hautes-Alpes, l'un des derniers départements desservis par un train de nuit, ce sujet me tient particulièrement à coeur et suscite bon nombre d'interrogations. Il faut dire que le Paris-Briançon fait figure de dinosaure tant il est resté depuis de nombreuses années en dehors de toute modernisation du réseau, en dehors de toute réflexion d'ensemble, qu'il s'agisse d'aménagement du territoire ou de moyen de transport sûr et efficient.

Le Paris-Cerbère, le Paris-Latour-de-Carol et le Paris-Briançon pourraient-ils finalement être les moyens les plus sûrs, les plus économiques et les plus écologiques de relier les territoires et la capitale ? Je le pense, et nous sommes d'ailleurs un certain nombre d'élus et d'usagers à partager ce point de vue. Pourtant, à ce stade, difficile d'être audible quand chaque passager coûte à l'État, quand le modèle économique est obsolète, quand le matériel roulant est inadapté, quand la fréquence est aléatoire et quand l'ouverture à la réservation se fait parfois de plus en plus tard. La SNCF voudrait dissuader les usagers des trains de nuit Intercités qu'elle ne s'y prendrait pas autrement ! Pourtant, force est de constater que ces trains affichent souvent complet, notamment le week-end et en période de vacances scolaires, par exemple. Ils correspondent à un certain type de clientèle. Si, sur d'autres périodes, les Intercités de nuit sont moins fréquentés, c'est que l'offre pourrait sans doute être améliorée. À l'heure des mouvements en faveur du climat et des initiatives pour limiter l'usage du transport aérien, responsable, je vous le rappelle, de 10 % des émissions de gaz à effet de serre, je n'ai pas senti de réelle volonté d'inscrire les trains de nuit dans la durée, au-delà du sursis de dix ans qui a été annoncé. Ils sont maintenus, faute d'alternative, mais ne bénéficient pas d'un engouement de la part de la puissance publique. Par exemple, en 2021, le Paris-Briançon sera remplacé par des autocars pendant plus de six mois, alors qu'un itinéraire de substitution aurait pu être envisagé s'il avait été jugé prioritaire. Mais, entre l'État, les régions et SNCF Réseau, la coordination est parfois délicate. Je déplore cette situation, vécue localement comme une véritable injustice. S'agissant des auto-trains, de nombreuses destinations ont été fermées faute d'un modèle économique adapté et, surtout, faute d'une volonté de mettre sur les rails des centaines de véhicules plutôt que d'encombrer les routes et de mettre des actes en adéquation avec des déclarations. En préparant mon intervention, j'ai tenté à plusieurs reprises de simuler un auto-train vers les gares qui apparaissaient comme desservies. Eh bien, c'est impossible ! La SNCF me propose des chauffeurs, des camions, mais aucun train ! train ! Des wagons porte-automobiles ne pourraient-ils pas être associés aux trains de nuit pour rétablir ce service de fret ? Des solutions techniques existent. J'ai rencontré récemment un porteur de projet d'une navette ferroviaire autonome qui pourrait répondre aux besoins des lignes d'importance locale. L'État a perdu la main en matière ferroviaire, comme le prouvent ses tergiversations sur l'étoile ferroviaire de Veynes et son incapacité à faire plier SNCF Réseau.

La SNCF, pour sa survie, s'est spécialisée sur le voyageur, la grande vitesse et le périurbain, privilégiant les secteurs où le transport peut être massifié. La SNCF, pour sa survie, a aussi tué, en plus des trains de nuit, les Intercités, le fret, les petites lignes.

a été contrainte de faire des économies importantes sur l'état du réseau, au prix de la sécurité. Le ferroviaire est une industrie de réseaux, avec un coût de création de l'infrastructure absolument

ÖBB, qui a réussi à conceptualiser une offre internationale, moderne, avec un modèle économique apparemment profitable. Regardons aussi la Suède, l'Écosse ou nos voisins suisses, exemplaires du point de vue ferroviaire.

l'un des objectifs du plan Massif central envisagé par Valéry Giscard d'Estaing en 1975 consistait en un désenclavement de la région. Las, nous

deux trains de nuit pour Paris par Brive et Clermont-Ferrand et deux trains directs vers Paris, ainsi que des trains de neige au départ de Périgueux, Brive, Limoges et Cosne-Cours-sur-Loire.

et seulement un train de neige au départ de Brive. La dégradation de la qualité du service sur la liaison Paris-Aurillac est particulièrement représentative du long désengagement de l'État concernant l'entretien des infrastructures ferroviaires existantes.

En 2003, le gouvernement Raffarin a supprimé les trains de nuit, qui permettaient encore d'effectuer l'aller-retour en une journée. L'année suivante, tous les trains directs entre Paris et Aurillac ont également été supprimés. Dès lors, dans ce cas de figure, le droit à la mobilité se résume à une offre ferroviaire défaillante, une première autoroute à près d'une heure trente du chef-lieu du Cantal,

En 2000, la SNCF a supprimé 300 points d'arrêts sur les soixante-sept trains de nuit qui circulaient encore tous les jours. L'abandon par l'État et la SNCF SNCF de l'ambition que l'on pouvait porter pour nos territoires a frappé l'ensemble des trains d'équilibre du territoire (TET), mais aussi d'autres petites lignes. Il a éteint les espoirs de nos concitoyens, qui ne peuvent se satisfaire de logiques comptables. Ce « recentrage » de l'offre, pour parler en langage technocratique, sur les derniers trains d'équilibre du territoire considérés comme structurants est mortifère pour la ruralité. Huit seulement ont été préservés, dont deux trains de nuit, d'autres lignes seront reprises par les régions, sans que l'on sache pour Leur fréquentation avait certes baissé et l'insuffisante rentabilité constituait l'excuse parfaite à ce sabotage. Encore fallait-il se pencher sur la véritable cause : le manque d'investissements consacrés aux infrastructures causait de multiples retards, décourageant, une fois de plus, les voyageurs. Tous gouvernements confondus, ces décisions laissent un goût amer à la ruralité, qui ressent une volonté de délaisser les liaisons peu rentables, les amenant à l'agonie pour provoquer leur fermeture. En ce qui concerne les auto-trains, après une réduction progressive de l'offre- cela débute toujours ainsi -, la SNCF prévoit déjà leur suppression d'ici à la fin de l'année, sans l'annoncer explicitement sur le site de réservation, tout en proposant le recours à un chauffeur. Je m'interroge sur les vertus écologiques de cette décision. Lors de la publication du rapport que j'ai commis, relatif à la contribution du transport aérien au désenclavement et à la cohésion des territoires, il m'a été reproché de faire la promotion de l'aérien au détriment des autres modes de transport. C'est méconnaître la réalité de l'enclavement, ainsi que mes engagements en faveur du retour de nos dessertes ferroviaires, qui restent prioritaires. Ce sont les fermetures successives des lignes de train vers les grandes villes que compte notre pays, ainsi que la dégradation de celles qui subsistaient, qui ont rendu vital le recours à l'avion. Pour certains endroits de notre pays, face à une demande de mobilité existante et une offre maigre, que ce soit à titre personnel ou professionnel, la seule réponse est la diversification de l'offre ferroviaire. C'est la raison pour laquelle, bien que cela ne soit pas dans l'air du temps, je souscris aux propositions de nos collègues visant à promouvoir l'auto-train et les trains de nuit. En l'absence de maintien de ces services, c'est le report du train vers la route ou l'avion qui est soutenu, pour ceux qui pourront encore se déplacer. L'urgence climatique implique un recours accru à des moyens de transport moins émetteurs de gaz à effet de serre, mais elle requiert plus d'équité pour rassembler efficacement, car la ruralité adhère à nos objectifs environnementaux si on lui donne la possibilité d'opérer la transition. N'opposons pas les moyens de transport lorsqu'il ne peut y avoir de report modal en l'état actuel des infrastructures ferroviaires. En ce qui concerne le mode aérien, sa transition écologique doit également être accompagnée. Le groupe du RDSE ne peut qu'apporter son soutien aux auteurs du débat, bien qu'il ne s'agisse que d'une partie de la réponse à un problème bien plus large, celui du droit à la mobilité et à un aménagement très équilibré de notre territoire. La parole est à M. Frédéric Marchand.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, notre débat de ce soir est, une fois encore, l'illustration que chemin de fer et récit national sont intimement liés. Le rail a apporté une contribution éclatante à l'aménagement de notre territoire national, du nord au sud et de l'est à l'ouest. En 2017, en lançant les Assises de la mobilité, le Gouvernement a initié une refonte sans précédent de la politique des transports avec l'objectif d'améliorer la mobilité de tous les Français, sur tous les territoires. Ces assises se sont prolongées l'an dernier par l'examen de la loi d'orientation des mobilités. Il a donné lieu, dans cet hémicycle, à des débats riches, sans tabou, visant une seule et même priorité : la mise en place d'un modèle, d'un cercle vertueux profitable aux usagers, aux entreprises ferroviaires, à l'État, aux collectivités territoriales et à l'aménagement du territoire et, surtout et encore, à la transition écologique. Nous prolongeons aujourd'hui ce débat autour de la situation des trains de nuit et de l'auto-train. les trains Intercités sont une catégorie résiduelle, entre grande vitesse et transport express régional. En effet, ces trains ne sont pas des TGV, car ils ne dépassent pas 200 km/h et circulent sur le réseau classique. Assurant des relations de moyenne et longue distance, ils ne sont pas non plus des TER, lesquels sont en principe chargés des dessertes locales dans le périmètre d'une région. le périmètre d'une région. Leur périmètre n'a cessé de se réduire, à la mesure du développement des deux autres activités. C'est d'abord la conséquence du développement du réseau à grande vitesse, qui, depuis une trentaine d'années, a peu à peu dominé la stratégie de la SNCF en matière de grandes lignes, concentrant, en ce domaine, les investissements en infrastructures, en matériel roulant, en stratégie commerciale et d'image. Toutefois, cette marginalisation est aussi à mettre en regard du développement du transport régional, qui, depuis une dizaine d'années, bénéficie pour sa part de l'implication des autorités organisatrices régionales et de leurs investissements. Circulant à la fois sur le réseau des grandes lignes et sur des portions du réseau ferré d'intérêt local, les trains Intercités doivent s'adapter à leurs disparités d'électrification : dix-huit lignes, soit plus de la moitié de celles qu'ils empruntent, ne sont que partiellement, voire pas du tout électrifiées. Enfin, les trains Intercités sont particulièrement touchés par le retard de rénovation du réseau ferré classique, qui a longtemps pâti de l'allocation prioritaire des investissements aux projets de lignes nouvelles à grande vitesse. Ces éléments font que les trains Intercités ont aujourd'hui une fréquentation globalement faible, avec un parc de trains assez obsolète. Il résulte de tous ces écueils que l'activité Intercités, de jour comme de nuit, n'occupe qu'une place minoritaire par rapport aux autres activités de transport de voyageurs de la SNCF. Elle est de plus en plus fortement concurrencée par le développement croissant des voyages et par de nouvelles solutions de covoiturage.

: il ne répondait plus aux besoins des voyageurs, engendrant de fait une forte baisse de la fréquentation et une augmentation importante du déficit financier. Ainsi, le gouvernement précédent a fait le choix d'un recentrage de l'offre de TET de nuit sur les lignes dont le caractère d'aménagement du territoire a été jugé essentiel au regard des populations desservies et du manque ou de l'absence d'une offre de transport alternative. En septembre 2018, lors d'un déplacement en train de nuit dans les Hautes-Alpes, la ministre Élisabeth Borne a réaffirmé que le train de nuit a un avenir, car il constitue une bonne solution pour l'accessibilité des territoires et un atout pour le développement économique et touristique. Elle s'est engagée pour la pérennité des deux lignes de nuit existantes, dont la convention d'exploitation sera reconduite au-delà de 2020 et dont on rénovera le matériel pour assurer la robustesse et la sécurité des rames, mais également pour répondre aux demandes légitimes des voyageurs quant à l'amélioration du confort.

Il peut donc être utile de reconsidérer les conclusions de la commission Duron sur l'avenir des trains d'équilibre du territoire, remises en 2015, et d'éclairer, dans ce nouveau contexte, les enjeux et les conditions d'un développement plus important du réseau des lignes de nuit, en cohérence avec le calendrier des travaux de remise en état de l'infrastructure. Par ailleurs, avec l'avènement d'une catégorie de touristes écoresponsables, on peut imaginer qu'au niveau européen le train de nuit soit envisagé comme une solution de substitution à l'avion. Abandonné un peu partout en Europe ces dernières années, le train de nuit transfrontalier renaît en Autriche : la compagnie nationale ÖBB développe son réseau depuis 2016. Elle est désormais leader dans l'offre de trains de nuit à travers l'Europe, avec vingt-six lignes, qu'elle opère seule ou en partenariat. Voilà un exemple qu'il serait bon d'étudier finement. Le Gouvernement propose de remettre un rapport au Parlement d'ici au 30 juin 2020, en s'inspirant notamment des expériences conduites dans d'autres pays pour imaginer un avenir aux trains de nuit. Cette annonce va bien entendu dans le bon sens. Le service auto-train, proposé par SNCF Mobilités, présente des avantages sur le plan environnemental et en termes de sécurité routière. Toutefois, ce service, qui s'appuyait initialement sur la circulation des trains de nuit, a connu une baisse d'activité considérable depuis une quarantaine d'années. Cette lente agonie a commencé au début des années 1980 avec le développement des autoroutes. Ainsi, en trente ans, le service a perdu 80 % de trafic et son modèle a largement évolué avec la disparition des trains auto-couchettes. L'érosion progressive du trafic est également liée au développement de la grande vitesse ferroviaire, qui a considérablement renforcé l'intérêt du train par rapport à la voiture pour les destinations desservies par TGV. Cette tendance s'est confirmée au cours des quatre dernières années, qu'il s'agisse du chiffre d'affaires ou du nombre de véhicules transportés, avec une diminution d'activité de 13 % depuis 2013. Une augmentation des prix a été effectuée, mais elle s'est révélée largement insuffisante pour redresser la situation économique de ce service, qui est aujourd'hui fortement déficitaire. En 2016, l'auto-train a perdu un peu moins de 10 millions d'euros, soit l'équivalent de son chiffre d'affaires. Les charges se rapportant à ce service sont, en effet, fixes pour les trois quarts d'entre elles, alors que l'activité est d'ores et déjà très saisonnière- elle se concentre à 70 % entre juin et septembre. SNCF Mobilités a donc décidé de restreindre le service aux destinations les plus demandées, soit Avignon, Marseille, Toulon, Fréjus et Nice. La situation de l'auto-train, certes dans le cas d'un marché de niche, illustre les enjeux environnementaux et les contraintes financières du transport ferroviaire. Pour remplacer ce service de transport de voitures par train, la SNCF train, la SNCF entend réorienter ses clients vers un concurrent, une start-up qui propose d'acheminer la voiture jusqu'à son lieu de destination de trois manières différentes : par un conducteur particulier, par un professionnel ou en camion.

pour le rendre à la fois économiquement efficace, plus performant en matière de qualité de service et essentiel à la réalisation de la transition écologique. En définitive, nous sommes arrivés à la fin d'un cycle, à la fin de la lente agonie des auto-trains : même

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, avec ce débat, les élus de mon groupe persistent et signent dans leur volonté de porter haut et fort le combat pour le redéploiement des trains de nuit. Il m'est difficile d'intervenir après le très riche propos liminaire de ma présidente de groupe, mais je vais tenter l'exercice Je ne développerai pas davantage l'incohérence totale de notre politique des transports, qui favorise encore et toujours la route et l'aérien au détriment du rail tout en prétendant vouloir agir contre le réchauffement climatique et la pollution. J'ajouterai deux arguments pour insister sur le bien-fondé d'une nouvelle offre de trains de nuit. Mon premier argument est que le train de nuit représente une offre de transport qui n'a pas de concurrence sur les longues distances. Aucune autre offre ne permet à un travailleur résidant dans le sud de la France et travaillant en région parisienne de passer une soirée avec sa famille avant de prendre son train et d'arriver sur son lieu de travail tôt le matin. Les derniers trains, les derniers avions du soir partent entre vingt heures et vingt et une heures ; les premiers trains ne permettent pas d'arriver à huit heures sur son lieu de travail, pas plus que les premiers avions, qui ne décollent pas avant six heures du matin. Pour tous ces travailleurs, la suppression des trains de nuit signifie, ou signifierait, une vie de famille amputée de précieux moments. Puisque nous parlons des travailleurs, je rappelle que dix millions d'entre eux sont en horaires décalés, dont une grande partie travaille de nuit. Pour tous ces travailleurs, le train de nuit et ses dessertes fines des territoires peuvent représenter une solution de substitution bienvenue et sécurisante par rapport à la voiture.

ce que nos amis Suédois, précurseurs en la matière, appellent le. On les comprend : le bilan carbone du secteur aérien est absolument désastreux. Je rappelle que, pour chaque kilomètre que vous faites en avion, vous émettez autant de CO2 que si vous parcouriez la même distance tout seul dans un petit camion. L'Allemagne, qui augmente les taxes sur l'avion en réduisant la TVA sur le ferroviaire, nous montre l'exemple à suivre pour corriger cette erreur. Cette honte de prendre l'avion est particulièrement prégnante dans la jeune génération, particulièrement sensible aux enjeux climatiques. Pour autant, cette génération est désireuse de voir le monde et, pour partie, elle entretient un rapport différent au voyage. Elle voyage en prenant le temps, en considérant le déplacement comme une part entière du voyage et non comme une translation entre un point de départ et un point d'arrivée. Cette forme de tourisme et de déplacement, qui tente de respecter au maximum notre environnement, doit être encouragée. Un élan européen de renaissance du train de nuit commence à poindre, en Suède, en Allemagne, en Autriche notamment. Monsieur le secrétaire d'État, nous vous invitons à porter ce dossier à Bruxelles, à vous coordonner avec nos voisins pour renforcer l'offre intereuropéenne de trains de nuit. Voilà une colonne vertébrale pour renforcer l'offre et assurer une solution alternative à l'avion l'avion ! À ce titre, le Gouvernement a promis 30 millions d'euros dans le budget pour 2020. C'est un premier pas bienvenu, mais qui demeure insuffisant pour développer une offre digne de ce nom, notamment aux deux extrémités du spectre voyageur l'offre de sièges inclinables pour les voyageurs les plus modestes et l'offre de cabines individuelles avec salle de bains pour les voyageurs professionnels pris en charge par leur entreprise. Parmi les points de détail, j'attire votre vigilance sur l'indigence des offres en ligne de la SNCF : de manière incompréhensible, les trains de nuit n'y sont souvent pas indiqués. Malgré tous ces handicaps, les trains de nuit qui subsistent en France ont un taux d'occupation de 45 % à 50 %, ce qui est remarquable. Le modèle autrichien nous montre que le seuil de rentabilité des trains de nuit se situe autour d'un taux d'occupation de 60 % ; l'effort à fournir pour y parvenir n'est donc pas énorme. autre aberration doit être corrigée pour développer le train de nuit : elle concerne les droits de péage des petites gares. Aujourd'hui, le train de nuit paie des péages dans chaque gare qu'il dessert. Cette situation n'incite pas à multiplier les arrêts, lesquels sont pourtant indispensables à son bon fonctionnement et à une desserte fine du territoire. Aujourd'hui, la gare d'Austerlitz est la gare la plus chère de France, alors qu'elle accueille beaucoup moins de trains que les autres gares parisiennes. C'est aberrant ! L'État doit inciter SNCF Réseau à déployer une tarification beaucoup plus incitative, voire à proposer un péage inversé, une sorte de bonus « aménagement du territoire

Je me réjouis naturellement de l'intérêt que vous portez à cette ligne- nous en avons déjà parlé -, dont je ne doute pas un instant de l'utilité. Vous le savez, cette option implique d'engager sans tarder les travaux de rénovation de l'étoile ferroviaire de Veynes, pour lesquels le Gouvernement a promis son concours financier.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, l'urgence peut-elle nous imposer la lenteur ? C'est une vraie question. Le climat est en danger, et c'est peut-être par des déplacements en trains qui ne roulent pas à grande vitesse que nous pourrions contribuer à le préserver. C'est en tout cas la réflexion à laquelle nous invite ce débat. « Prenez le temps d'aller vite », nous disait la SNCF en faisant la promotion du TGV. Il s'agit effectivement d'une prouesse technologique que le monde nous envie. Le TGV a permis de raccourcir les distances comme jamais : Marseille est à trois heures quinze de Avons-nous cependant toujours besoin d'aller si vite ? Le TGV remplit bien sûr un besoin existant, mais est-il systématiquement nécessaire ? « Le train, l'automobile du pauvre. Il ne lui manque que de pouvoir aller partout », écrivait Jules Renard. La pertinence de ces mots a évolué avec le temps. Son prix a augmenté, mais le train continue de ne pas aller partout : il dessert même de moins en moins de lieux, car, pour aller vite, il n'est pas possible de s'arrêter dans toutes les gares. Il existe pourtant tout un monde entre les grandes villes françaises. Ce monde, par définition, ne peut pas être desservi par le TGV. Nos territoires ont besoin, en plus des lignes à grande vitesse, de lignes de desserte fine pour permettre à tous de se déplacer. Nous avons besoin d'avoir le choix. pourraient utilement compléter l'offre actuelle. Ils ont le double avantage de desservir plus de gares et de rendre les longs trajets plus agréables et plus commodes.

Ce dernier était, hélas ! insuffisamment connu de nos concitoyens. C'est peut-être pourquoi il n'était pas assez utilisé, alors même qu'il a toute sa place dans le panel des modes de transport. Sa disparition a entraîné une hausse de l'utilisation des automobiles et, donc, des conséquences écologiques négatives. Nous ne devons pas nous restreindre à une alternative opposant le TGV au transport routier. C'est pourtant ce que semblent privilégier certains en prônant l'interdiction des vols intérieurs. chaque mode de transport a son utilité. Nous sommes convaincus que les usagers doivent avoir le choix. Nous sommes également convaincus que le prix des voyages doit refléter l'impact écologique, afin que les moins polluants soient les moins chers. Le train est un moyen de transport d'avenir. De nouvelles technologies sont à l'étude, comme le train à hydrogène : la SNCF a annoncé que les premiers trains de ce type circuleraient en France d'ici à deux ans. il a beaucoup été question des trains légers, qui sont susceptibles de faire évoluer le seuil de rentabilité des voyages ferroviaires. Le transport ferroviaire doit continuer de se verdir. En ce sens, nous souhaitons que les services d'auto-train et les trains de nuit puissent de nouveau circuler en France. Pour paraphraser la SNCF,

le train de nuit revient à la mode, paraît-il ... Moins polluant que les autres moyens de transport et plus sûr que la voiture ou le bus, il présente beaucoup d'avantages pour des trajets de des trajets de longue distance. Pourtant, nous sommes quelques-uns ici à pouvoir en témoigner, il y a à peine deux ans, nous redoutions sa suppression définitive. notre crainte à la ministre, Mme Borne, et elle s'était engagée à maintenir les deux lignes restantes, dont le Paris-Rodez, qui concerne mon département de l'Aveyron. Cette ligne de train de nuit est notre seule liaison directe terrestre avec Paris. Comme beaucoup d'autres lignes de nuit desservant les villes moyennes, les Millau-Paris et les Villefranche-de-Rouergue-Paris ont été supprimés. Les conséquences sur l'attractivité de ces territoires sont bien visibles. Le train de nuit Paris-Rodez a, lui aussi, failli disparaître ; si elle n'a pas encore disparu, cette liaison est en grande souffrance. La politique du tout-TGV n'a rien laissé aux trains de nuit.

Malgré toutes ces difficultés, le taux de remplissage du Paris-Rodez avoisine les 50 %. Oui, pour nous, Aveyronnais, le train de nuit présente de nombreux avantages ! Il est utilisé depuis longtemps par toutes les générations. Il est le moyen de transport le plus facile et le moins cher pour monter à Paris ou pour descendre au pays. La liaison est directe. On arrive ici en centre-ville, sans être coincé dans les nombreux embouteillages. On ne perd pas une demi-journée ou une journée dans la voiture ou du fait des nombreuses correspondances en passant par Toulouse, Montpellier ou Clermont-Ferrand.

il devient urgent, comme l'Autriche et la Suède viennent de le faire, de réinvestir dans les trains de nuit et de les promouvoir. On pourrait rouvrir d'anciennes lignes ou imaginer de nouveaux itinéraires en France ou vers l'étranger. Il est plus que nécessaire de moderniser ces trains et d'assurer un niveau suffisant de confort, qu'il s'agisse des sièges inclinables- M. Gontard vient de le rappeler -ou des couchettes. Une nouvelle clientèle est prête à s'approprier le train de nuit : la demande est là, mais l'offre n'existe pas ou n'est pas adaptée.

sans doute à des destinations plus touristiques ou à de plus grandes villes, notre train de nuit Paris-Rodez ne serait plus menacé comme il l'a été durant tant d'années. d'années. En somme, par leurs pratiques et par leur attachement au train de nuit, les Aveyronnais, que je représente ici, faisaient de l'écologie avant la prise de conscience de l'urgence climatique qui est aujourd'hui d'actualité.

Jamais l'État n'a fait un diagnostic complet et apporté une réponse globale aux problèmes du ferroviaire. [ ...] La vraie casse du service public, c'est quand on a près de 20 % des lignes qui sont ralenties par manque d'entretien comme aujourd'hui. La vraie casse du service public, c'est quand on laisse se dégrader la qualité du service dans les trains de nuit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de voyageurs et qu'on arrête ces trains. La casse du service public, c'est de laisser perdurer la situation actuelle Ces mots ne sont pas ceux d'un syndicat du rail, mais ceux d'Élisabeth Borne dans une interview accordée au en février 2018. En tant que rapporteur spécial du budget des transports, j'approuve ce constat. Il est effectivement urgent d'agir : urgent d'agir pour financer la régénération ferroviaire, urgent d'agir pour moderniser notre aiguillage. Toutefois, au-delà des trains de nuit et des auto-trains, il me semble nécessaire d'élargir le débat pour parler des trains de fret. Les besoins de transports liés au développement économique devraient augmenter de 30 % à horizon de 2030. À parts modales inchangées, l'augmentation des émissions de CO2 serait alors de 80 millions de tonnes par an. Le ferroviaire a toute sa place dans la transition écologique à laquelle aspirent nos concitoyens. Aujourd'hui, le transport ferroviaire représente seulement 11 % du transport intérieur de passagers et à peine 10 % du transport intérieur Pourtant, un train de fret émet seulement 3 tonnes de CO2 et permet d'éviter quarante-cinq poids lourds sur la route, qui, cumulés, représenteraient 44 tonnes de CO2.

Très exposées à la conjoncture économique, souffrant de la concurrence routière sur un marché tout de même relativement étroit, les entreprises de fret ferroviaire connaissent toutes des difficultés économiques.

Deuxièmement, l'État compte-t-il abandonner aux régions la gestion des lignes capillaires de fret ? Si oui, avec quels moyens ? Très récemment, la région Hauts-de-France est venue en soutien à deux lignes qui auraient dû fermer : la ligne Valenciennes-Quiévrain et la ligne Compiègne-Lamotte-Breuil.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, nombreux sont les débats qui ont eu lieu dans cet hémicycle à propos du transport ferroviaire. Malheureusement, nous dressons toujours le même constat : une offre de service public qui diminue, des infrastructures qui manquent d'investissements et, surtout, un secteur qui souffre face à la concurrence de l'aérien et du routier. La récente annonce de la suppression des auto-trains en est un exemple supplémentaire. La SNCF se justifie en indiquant que le service est structurellement déficitaire à cause du faible remplissage de ces trains, ce qui entraîne une perte de chiffre d'affaires. Mais il est difficile de se satisfaire d'un argument comptable. Dans quelques jours, l'auto-train sera remplacé par une start-up qui propose l'acheminement par un chauffeur particulier ou par un professionnel.

Ne faudrait-il pas imaginer d'autres solutions ou remettre au goût du jour des services qui ont existé, mais qui, faute d'avoir pu évoluer, ont disparu alors même qu'ils présentent de nombreux avantages ? Je pense bien sûr aux trains de nuit. Il est indéniable que ce service devait se réformer et que des améliorations étaient nécessaires ; les trains de nuit présentent néanmoins une double pertinence pour l'aménagement du territoire et pour la revitalisation des centres.

En l'absence d'une telle offre, les villes moyennes éloignées les unes des autres sont mal connectées entre elles. En effet, les liaisons aériennes entre deux villes moyennes sont rares et onéreuses. En effectuant ces trajets de nuit,

début 2022. En Suisse, le trafic de nuit a augmenté de 25 % depuis le début de Le train de nuit peut également être un complément efficient aux lignes à grande vitesse et pourrait présenter une offre de mobilité touristique attractive. Pour cela, il faudrait bien sûr investir davantage : les 30 millions d'euros promis par le Gouvernement sont loin d'être satisfaisants, sachant que, parmi les différents scenarii proposés par la SNCF, on a choisi l'enveloppe minimale, permettant tout juste de rénover le nombre suffisant de voitures. Par ailleurs, il faudrait réfléchir à l'articulation entre l'organisation du trafic et les nombreux travaux engagés sur les voies, qui s'effectuent essentiellement de nuit.

De manière générale, pour optimiser les mobilités, ne faudrait-il pas favoriser les trains mixtes, comme les trains auto-couchettes ou les trains de nuit voyageurs-marchandises ?

L'offre de transports publics doit répondre aux différents besoins, qu'il s'agisse des citoyens ou des collectivités, tout en permettant à chacun de se déplacer de manière écologiquement responsable. La parole est

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, que de temps perdu ! Alors qu'en 2016 l'État annonçait la suppression de la totalité des trains de nuit, rebasculant ainsi une partie du trafic ferroviaire sur la route les solutions de covoiturage ou les cars Macron, la priorité qui taraude la Commission européenne, et à laquelle je souscris pleinement, est bien de savoir comment transférer les passagers de la route vers le rail afin de réduire les émissions polluantes. Si les émissions du secteur des transports représentent actuellement plus d'un quart de l'empreinte carbone totale de l'Union européenne, le train, lui, ne représente que 3 % de ces émissions, quand la route est responsable de plus de 70 %. Or la Commission, qui devrait prochainement présenter un, a identifié les difficultés qui pourraient contrecarrer l'objectif d'un continent neutre en carbone d'ici à 2050. La première concerne l'état des infrastructures. En effet, l'objectif de l'Union est de transférer 30 % du transport routier effectuant des distances de plus de 300 kilomètres vers le train et les barges d'ici à 2030 et d'atteindre 50 % d'ici à 2050. Or les infrastructures ferroviaires ne peuvent, en l'état actuel, répondre à une telle hausse du trafic. La preuve en est que, en Allemagne, un train de longue distance sur quatre est maintenant retardé, en partie en raison des problèmes de capacité du réseau ferroviaire allemand. De même, dans leur majorité, les grandes villes sont en difficulté, car les hubs importants tournent à pleine capacité. Une première réponse consisterait donc à promouvoir les auto-trains et les Intercités de nuit, à l'heure où la demande est croissante, sous l'effet cumulé du prix élevé des billets de TGV et d'une certaine culpabilité

ces solutions sera, à court terme, d'utiliser le potentiel de capacité des infrastructures, notamment la nuit. La seconde difficulté identifiée par la Commission européenne concerne les financements. La suppression de trains Intercités et de trains de nuit a été, en 2016, le résultat malheureux de l'abandon de l'écotaxe, laquelle devait alimenter le budget de l'Agence de financement des infrastructures de Cet abandon a été à l'origine d'un manque à gagner terrible pour l'État, au détriment de plus de soixante lignes de trains de nuit qui se déployaient alors sur le territoire français. Dès lors, il nous faut nous donner les moyens de réinvestir dans le rail. Il est ainsi estimé que quelque 500 milliards d'euros seront nécessaires d'ici à 2030 pour achever les travaux sur les réseaux ferrés transeuropéens.

Au niveau national, vous n'êtes pas sans savoir que la loi d'orientation des mobilités n'est pas à la hauteur des enjeux ferroviaires, en raison d'une programmation au rabais des investissements de l'État dans les transports pour les dix prochaines années

Le ferroviaire constitue donc une véritable solution pour répondre au défi climatique. Nous en sommes tous ici convaincus. J'ajoute qu'il représente également un véritable enjeu d'aménagement du territoire : la promotion

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, ce débat est placé sous l'angle du rapport entre le ferroviaire, plus particulièrement les auto-trains et les trains de nuit, et l'urgence climatique.

Reste que, loin de nos débats, loin de l'hémicycle, loin des grandes conférences internationales sur le climat, des décisions sont prises qui produisent souvent l'effet exactement inverse à ces grands engagements.

la fermeture de la ligne d'auto-train Paris-Biarritz aura remis chaque été plus de 20 000 véhicules sur les routes. Cette mesure va bien à l'encontre de la réduction de l'empreinte écologique. La suppression de nombreux trains de nuit est également allée à contresens des objectifs affichés. Pour sa défense, la direction de la SNCF a bien laissé entendre que ces trains de nuit étaient vides et que leur exploitation était déficitaire, mais l'Autorité de régulation des transports a rectifié le tir précisant que le taux d'occupation des trains de nuit était, en 2015, de près de 10 points au-dessus de la moyenne de l'activité des Intercités. Dans les Pyrénées-Atlantiques, département frontalier de l'Espagne, ces suppressions sont d'autant moins compréhensibles que l'ART avait relevé que la ligne Paris-Hendaye était l'une des plus performantes et présentait, par ailleurs, un fort potentiel de développement, avec la possibilité d'une liaison jusqu'à Irún permettant de rejoindre, à court terme, San Sebastián, puis d'autres villes espagnoles. De même, à propos de la célèbre Palombe bleue, le Président de la République n'avait-il pas déclaré, lors de son déplacement à Bagnères-de-Bigorre en juillet 2019 : « La Palombe, je l'ai prise plein de fois ! Il faudrait investir ici.

qui est aujourd'hui trop réduite en France. Je salue cette évolution qui, au-delà de ses objectifs écologiques, contribuera au développement des territoires. Toutefois, le flou demeure sur les moyens de faire revivre l'auto-train et les trains de nuit.

fort peu. Il sera tôt ou tard nécessaire de commander du matériel neuf, et cela prendra plusieurs années. En attendant, pour réduire les coûts de redémarrage des trains de nuit, il serait urgent de prendre des mesures conservatoires pour sauvegarder autant que possible une part plus importante du parc Corail existant. J'ai donc plusieurs questions. Pour les opérateurs entrants sur ce marché et qui manquent de matériel roulant, allez-vous formuler des propositions ?

Cela me donne l'occasion, au lendemain du vote définitif de la loi d'orientation des mobilités, de réaffirmer devant vous l'attachement profond du Gouvernement au transport ferroviaire. Il s'agit d'un mode peu polluant, rapide et sûr, dont nous souhaitons le développement au bénéfice de toutes les Françaises et de tous les Français sur l'ensemble du territoire national. À travers le nouveau pacte ferroviaire adopté en 2018, le Gouvernement est déterminé à réformer le système ferroviaire, pour le rendre plus performant pour les usagers et plus efficace sur le plan économique. Il s'agit de faire plus et mieux, avec une meilleure qualité de service et à moindre coût. Des marges de manoeuvre existent, et c'est en gagnant sur ces marges que nous pourrons atteindre nos objectifs en matière de transition écologique.

Faire plus et mieux dans le domaine ferroviaire, cela signifie accepter de faire évoluer ce service public, dans lequel l'histoire et la tradition pèsent particulièrement lourd. Cela pourra, et devra, passer par des transformations parfois difficiles, tant l'attachement des cheminots, des élus et des citoyens à ces services est profond. En tant que membre du Gouvernement, mon devoir est d'accompagner ces changements, en répondant aux craintes et à la nostalgie qui peuvent s'exprimer parfois à juste titre. Après ce propos liminaire, j'en viens au premier objet de notre débat : le service auto-train. Créé en 1957, il a connu une baisse d'activité considérable et continue depuis une quarantaine d'années. Malgré l'augmentation des prix réalisée par SNCF Mobilités il y a quelques années pour tenter de revenir à l'équilibre financier, le service est resté fortement déficitaire. En 2016 et 2017, il a ainsi perdu environ 10 millions d'euros, soit l'équivalent de son chiffre d'affaires. Dans ces conditions, SNCF Mobilités a décidé, en 2018, de le restreindre aux destinations les plus demandées : Avignon, Marseille, Toulon, Fréjus-Saint-Raphaël et Nice. Les résultats de 2019 confirment cette tendance, et le niveau de fréquentation devrait une nouvelle fois baisser pour atteindre moins de 29 000 véhicules transportés. Ce constat explique pourquoi SNCF Mobilités a pris la décision de mettre un terme à ce service en décembre 2019. Il s'agit d'un choix relevant de la liberté stratégique et commerciale de l'entreprise.

Par ailleurs, tous les usagers de l'auto-train ne seront pas contraints de se reporter vers la route. La loi d'orientation des mobilités, votée hier, permet en effet de démultiplier les solutions alternatives à l'automobile sur les territoires. Le développement de la grande vitesse ferroviaire, qui est une fierté nationale, et d'autres offres de mobilité, comme le recours accru aux alternatives à la voiture individuelle, ont significativement modifié les habitudes des Français depuis quarante ans. Ainsi, un voyage en auto-train peut aujourd'hui être avantageusement remplacé par un voyage en train de passagers, encore plus écologique, combiné avec une location de voiture en autopartage ou un trajet en covoiturage à l'arrivée. les nouvelles formes de mobilité nous invitent à revisiter notre rapport à la voiture individuelle, et l'auto-train était voué à un certain déclin au fur et à mesure que le rapport de nos concitoyens à la propriété de l'automobile évoluait. Le Gouvernement est attaché à ce que les services ferroviaires, quand ils répondent à un besoin, puissent trouver les conditions qui leur permettent d'atteindre l'équilibre d'exploitation. Ce n'est sans doute plus le cas du service auto-train, qui était utile à nos concitoyens à sa création et encore dans les années 1980, mais qui correspondait de moins en moins à leurs besoins. S'agissant du sujet des trains de nuit, la dynamique est très différente. Ce mode suscite un fort regain d'engouement depuis quelque temps. Pour commencer, j'aimerais rappeler l'historique récent de ce service et la logique qui a prévalu à la suppression d'un certain nombre de lignes. Ce rappel nous permettra d'aborder sereinement l'avenir pour bâtir des offres en mesure de satisfaire la demande des usagers pour le train de nuit, dont personne aujourd'hui ne conteste l'existence. En 2015, la commission « TET d'avenir », présidée par Philippe Duron, alors député, a démontré que l'offre de nuit telle qu'elle existait alors, faisant partie des trains d'équilibre du territoire, ne répondait plus de manière satisfaisante aux besoins des voyageurs et présentait un modèle économique très dégradé. Ces lignes se heurtaient alors à de fortes baisses de fréquentation, dues, notamment, au développement des vols intérieurs et de certains TGV, qui rendent possibles des départs tôt le matin et des retours tard le soir, ainsi que de la généralisation d'hébergements bon marché rendant compétitifs un déplacement de jour et une nuit sur place. Le précédent gouvernement a décidé, en 2015, d'arrêter progressivement le financement de ces lignes, à l'exception de deux lignes d'aménagement du territoire indispensables en raison de l'absence d'une offre alternative suffisante. Il s'agit des lignes de nuit desservant de nuit desservant depuis Paris Gap, Briançon, Rodez et Latour-de-Carol, circulant à raison d'un aller-retour quotidien. Toutefois, avant de prendre cette décision, l'État a souhaité tester les autres opérateurs ferroviaires, en les invitant à proposer, pour leur propre compte, de nouveaux schémas d'exploitation innovants. Un appel à manifestation d'intérêt a été lancé en 2016, mais aucune proposition pertinente n'a émergé. Le gouvernement précédent a donc maintenu sa décision de tarir le financement, restant à l'écoute de propositions qui émaneraient de collectivités territoriales. C'est dans ce cadre que la région Occitanie a montré son intérêt pour la réouverture de la desserte Perpignan-Cerbère. Un partenariat a été noué avec l'État pour la création, en juillet 2017, d'une nouvelle « antenne » au train descendant dans le sud-ouest afin de desservir les Pyrénées-Orientales le week-end et pendant les vacances scolaires de la zone francilienne.

J'aimerais désormais rappeler les annonces d'Élisabeth Borne, il y a maintenant un peu plus d'un an. Elle a déclaré que le train de nuit avait un avenir, car il constituait une solution adaptée pour l'accessibilité des territoires et un atout pour le développement économique et touristique. Elle s'est engagée sur la pérennité des deux lignes de nuit existantes, sur la reconduction de leur conventionnement au-delà de 2020 et sur la rénovation du matériel roulant pour un montant estimé aujourd'hui à 44 millions d'euros. C'est une première étape importante dans la reconsidération de ce moyen de transport et, là encore, un signe de la confiance du Gouvernement dans l'intérêt que représente le train de nuit. Je reprends cet engagement à mon compte, et je peux vous assurer qu'il sera tenu. Au-delà, je suis conscient que les préoccupations de la société, en particulier environnementales, modifient le contexte qui a prévalu jusqu'à présent et qui a permis le maintien d'un noyau de lignes très resserré au nom de l'aménagement du territoire. L'impératif écologique fait émerger de nouvelles perspectives économiques pour les trains de nuit. Les chiffres de fréquentation de l'année 2019 nous encouragent d'ailleurs dans cette voie, notamment chez nos voisins européens, où le train de nuit connaît souvent un franc succès. Pour ma part, je souhaite partager avec vous la conviction que le train de nuit peut constituer non seulement une offre de transport nécessaire pour répondre à des enjeux forts d'aménagement du territoire, du fait de l'absence d'alternative, mais aussi une offre écologique et sociale pour voyager sur de longues distances. Dans ce contexte, le rapport annexé à la LOM prévoit que, « d'ici au 30 juin 2020, l'État étudie également le développement de nouvelles lignes de TET, en veillant à son articulation avec le programme de régénération et de modernisation du réseau ferroviaire et en précisant, en particulier, les conditions d'une amélioration de l'offre des trains de nuit au regard de leur intérêt pour répondre aux besoins de désenclavement des territoires les plus éloignés des grands axes de circulation ainsi que de liaisons nationales et intraeuropéennes et pour réduire l'empreinte écologique. Cette étude est transmise au Parlement Cette étude est transmise au Parlement ». Je vous confirme que mes services travaillent d'ores et déjà sur cette étude. Je mesure l'attention qu'elle va concentrer, et je me tiendrai personnellement informé de son évolution au cours des prochains mois. L'une des principales problématiques est celle du matériel roulant, qui devra être renouvelé et donc faire l'objet d'un financement. Un certain nombre d'acteurs, aussi bien des élus que des associations, préconise de s'inspirer du réseau de trains de nuit élaboré par les chemins de fer autrichiens, ÖBB. En effet, ce réseau a repris un certain nombre de lignes de nuit délaissées par les réseaux limitrophes, en particulier en Allemagne. Cet exemple sera donc analysé finement dans le cadre de l'étude. Cependant, je tiens d'ores et déjà à appeler votre attention sur le fait que cet exemple ne peut être transposé tel quel au réseau français. Tout d'abord, les dessertes de nuit mises en oeuvre par ÖBB n'utilisent que des lignes électrifiées, ce qui permet des économies d'exploitation. Or la France comporte plusieurs territoires, comme l'Aveyron et les Hautes-Alpes, qui exigent des dessertes thermiques. Ensuite, la démographie de l'Europe centrale permet la mise en place de lignes reliant des agglomérations de plusieurs millions d'habitants entre Berlin, Prague, Budapest, ce qui n'est pas le cas chez nous, en raison d'une densité de population plus faible. Enfin, la France dispose d'un réseau de TGV beaucoup plus étoffé permettant d'offrir des dessertes de jour à longue distance plus efficaces que dans tout le reste de l'Europe. Il convient donc de considérer les bonnes pratiques qui pourront être transposées et de réfléchir à un nouveau modèle adapté à la France. Ces perspectives feront partie intégrante de la stratégie mise en place par l'État. Nous étudierons aussi les possibilités de développement du train de nuit à l'international. Il existe déjà un train reliant Paris aux métropoles italiennes de Milan et de Venise notamment. Le secteur privé ne manquera pas d'adapter d'adapter des services de qualité à une demande commerciale, et je compte bien accompagner favorablement ces démarches. Mesdames et messieurs les sénateurs, vous le voyez, le Gouvernement est résolument engagé pour l'avenir du train de nuit, qui s'inscrit dans sa politique, résolument tournée vers le ferroviaire en général.

Si l'on ajoute le budget de la LOM et celui des différents programmes budgétaires, 70 % des différents crédits sont donc alloués au mode ferroviaire. J'ai déjà eu l'occasion d'en produire le détail en commission, il y a quelques jours.

nous lions évidemment les travaux sur le Paris-Briançon à ceux qui sont actuellement à l'étude sur la ligne Nord-Sud entre Grenoble et Gap. À cet effet, la prochaine réunion copilotée par le préfet Dartout se tiendra le 4 décembre, dans le but d'aller vers une solution pérenne qui nous permette de solidifier ces deux axes, notamment l'axe de transport quotidien particulièrement important entre Grenoble et Gap.

S'agissant du fret, je lie ce sujet au travail important de régénération qui est déjà entrepris et qui va être encore

telle aviation. Dans une industrie de construction hautement capitalistique et aujourd'hui très largement duopolaire, pour utiliser un terme technocratique, nous pouvons envisager des perspectives tout à fait intéressantes en termes de croissance et d'emplois.